les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie mardi 9 avril sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement et du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai le grand plaisir de vous cet après-midi le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. La création de ce grand établissement

puisqu'elle recèle 10 % des espèces connues au niveau mondial, essentiellement grâce à nos outre-mer et à notre espace maritime. Mais cette biodiversité est en danger. Près de 30 % des espèces sont menacées ou quasi menacées sur notre territoire du fait d'activités humaines - pollutions, artificialisation des sols, fragmentation des habitats, surexploitation des espèces -et du développement d'espèces exotiques envahissantes. Pourtant, nous le savons, la biodiversité nous rend des services inestimables : les milieux humides nous fournissent l'eau potable, les insectes pollinisent nos cultures, les dunes et les mangroves nous protègent des tempêtes, les océans régulent le climat Le Gouvernement a donc lancé une action déterminée dans le domaine de la biodiversité. Cette reconquête passe par la création d'un opérateur de premier plan permettant d'appréhender tous les aspects de la biodiversité sur tous les types de milieux- terrestres, aquatiques, marins, y compris ultramarins

Je voudrais néanmoins revenir sur quelques points. Je commencerai par le nom de l'établissement. Le Gouvernement avait proposé- son amendement en ce sens avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale -de l'appeler « Office français de la biodiversité ». La commission a souhaité y ajouter le mot « chasse ».

Lors des discussions à l'Assemblée nationale, j'ai été amenée à donner un ordre de grandeur sur la taille de ce conseil, qui comprendra entre 30 et 40 membres. Les travaux préalables ont permis de préciser la représentation des parties prenantes, avec un conseil d'administration équilibré. Un comité d'orientation adossé à ce conseil d'administration aura vocation à être plus largement ouvert.

S'agissant d'un établissement public de l'État auquel sont confiées des missions régaliennes de police, le Gouvernement est attaché à conserver la majorité au conseil d'administration dans le premier collège, celui qui regroupe les représentants de l'État et les personnalités qualifiées. Afin de concilier une taille raisonnable du conseil d'administration, la diversité des parties prenantes et la nécessaire majorité accordée à l'État, le Gouvernement portera un amendement, que nous espérons de compromis, en vue de confier plusieurs voix aux administrateurs représentant l'État, donc de maîtriser la taille de cet organe.

pour sécuriser le budget de fonctionnement de l'établissement fusionné -et pour la contribution annoncée qui abondera la contribution des chasseurs aux actions concourant directement à la biodiversité. En effet, chaque chasseur financera à hauteur de 5 euros par permis de chasse une contribution qui sera abondée par la puissance publique à hauteur de 10 euros, laquelle, je le répète, sera également financée.

Je dirige personnellement son comité de pilotage, qui associe le « préfigurateur », les deux directeurs généraux de l'AFB et de l'ONCFS, les deux ministères qui concourent à la tutelle, les services déconcentrés du ministère de l'écologie et les agences de l'eau. Le dialogue social est également engagé avec les organisations syndicales, qui portent une demande légitime de requalification des inspecteurs de l'environnement de la catégorie C en catégorie B, et de reconnaissance plus grande des chefs de services départementaux.

mais une hausse des accidents avec blessés- 130, contre 113 lors de la saison précédente -et des incidents avec des dégâts matériels. Le projet de loi prévoit que l'accompagnateur d'un jeune chasseur devra suivre une formation spécifique. Nous souhaitons, en liaison avec le monde de la chasse, aller un peu plus loin. Le Gouvernement proposera donc deux amendements, qui tendent à prévoir, l'un des obligations minimales de sécurité pour homogénéiser les règles de sécurité à la chasse, l'autre, un dispositif de rétention-suspension du permis en cas d'accident ou d'incident matériel, sur le modèle du permis de conduire. Une autre question importante, dont nous aurons largement l'occasion de débattre, concerne les dégâts de gibier. L'enjeu est de mieux réguler le grand gibier, dont les populations s'accroissent fortement, afin d'enrayer l'augmentation des dégâts sur les cultures et les boisements. avant tout de prévenir et de développer une approche globale, ce à quoi invite le rapport de la mission parlementaire du député Alain Perea et de votre collègue Jean-Noël Cardoux, deux grands spécialistes du sujet.

prévues la responsabilisation financière des fédérations départementales dans l'indemnisation des dégâts, qui est souhaitée par la FNC et qui fait partie de l'équilibre de la réforme, la suppression de la péréquation financière directe au niveau national

Enfin, le projet de loi prévoit le transfert aux fédérations départementales de la gestion des associations communales de chasse agréées, les ACCA, et des plans de chasse, en leur donnant davantage de leviers pour agir. L'État interviendra en cas de défaillance grave des fédérations, et restera compétent pour fixer les objectifs de prélèvements d'espèces au niveau départemental. Ces transferts de mission seront compensés financièrement dans le cadre du financement global de la réforme. Cette réforme prévoit également la mise en place de la gestion adaptative des espèces. Une chasse plus durable permet de mieux adapter le niveau de prélèvement d'une espèce à son état de conservation. Un comité d'experts scientifiques a été créé au début du mois de mars pour faire des propositions en la matière. Le projet de loi précise la définition de cette gestion adaptative renvoie à un décret le soin de préciser la liste des espèces concernées. Il met en place une obligation de déclaration des prélèvements et la fixation de quotas de prélèvement pour les espèces concernées. Enfin, le projet de loi prévoit une contribution de 5 euros par permis de chasse et par an pour financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité. Le Gouvernement s'est engagé à soutenir ces actions à hauteur de 10 euros par an et par chasseur. La déclinaison des modalités de mobilisation de cette contrepartie fait l'objet d'un travail conjoint de l'AFB, l'ONCFS et la FNC, qui avance bien et qui devrait être formalisé sous la forme d'une convention-cadre nationale, à laquelle seront associées, en tant que de besoin, les agences de l'eau, afin que ces actions concourent directement à la biodiversité et financent des projets dans les territoires. Le Gouvernement présentera enfin un amendement visant à préciser l'organisation du Fichier national du permis de chasser, qui sera composé d'une base des permis délivrés alimentée par l'ONCFS, et bientôt par l'OFB, et d'une base des validations de permis gérée par la FNC et alimentée par les fédérations départementales. Ces deux bases sont, depuis très récemment, opérationnelles et interconnectées grâce à un travail conjoint, que je salue, mené par les fédérations de chasseurs, l'ONCFS et l'AFB. Le troisième Le troisième volet de ce texte renforce la police de l'environnement, sous ses deux aspects de police judiciaire et de police administrative. Pour la police judiciaire, le projet de loi procède à une extension significative des prérogatives des inspecteurs de l'environnement pour leur permettre de mener des enquêtes ordinaires ordinaires en totalité, de la constatation de l'infraction jusqu'à l'orientation de poursuites une fois l'enquête achevée, sans qu'il y ait lieu de se dessaisir au profit d'un officier de police judiciaire,

Une mission sur la justice environnementale a par ailleurs été engagée conjointement par la chancellerie et par le ministère de la transition écologique et solidaire. Elle a identifié quelques évolutions utiles, qui conduisent le Gouvernement à proposer des amendements. mission ne recommande pas à ce stade d'affecter aux inspecteurs de l'environnement des pouvoirs de coercition, du type garde à vue, seule prérogative qui distinguera encore les inspecteurs de l'environnement des OPJ au regard des nouveaux pouvoirs qui leur seront conférés.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues,près de trois ans après l'adoption de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, nous examinons aujourd'hui le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, ainsi qu'un projet de loi organique complémentaire, portant sur l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Permettez-moi de rappeler que la loi biodiversité de 2016 a permis la création de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, à partir du regroupement de quatre organismes publics l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'Onema, Parcs nationaux de France, l'Agence des aires marines protégées et l'Atelier technique des espaces naturels, L'objectif était alors de rassembler les opérateurs de l'État actifs en matière de biodiversité dans une seule et même entité, afin de simplifier et de renforcer les actions menées par l'État dans ce domaine. Lors de l'examen du projet de loi « biodiversité » en 2016, il était peut-être prématuré d'y intégrer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ONCFS. Ce délai supplémentaire a permis de poursuivre les échanges avec les parties prenantes, pour envisager aujourd'hui un rapprochement apaisé entre l'AFB et l'ONCFS. De ce projet de réforme, nous partageons les principales orientations et dispositions, à savoir la mise en place d'un nouvel établissement public, le renforcement de la police de l'environnement et une responsabilisation accrue des acteurs du monde de la chasse en faveur de la biodiversité. Il faut le rappeler, les chasseurs sont les premiers observateurs au quotidien de la biodiversité. Ils arpentent de long en large nos différents territoires. Ils sont les premiers à constater les changements de la nature ou les dépôts sauvages, par exemple. Dans certains territoires, la nature est rude, voire hostile. Elle a besoin d'être entretenue pour offrir les paysages époustouflants qu'admirent les nombreux touristes l'été. Les chasseurs contribuent bénévolement à la mise en valeur de cette biodiversité, à laquelle ils sont très attachés. Néanmoins, le texte transmis par l'Assemblée nationale présentait certaines lacunes, qui appelaient des clarifications et un rééquilibrage général, en vue de répondre à des inquiétudes persistantes sur ce projet de fusion.

d'études Chasse et pêche, avec lequel nous nous sommes constamment concertés pour élaborer un texte riche et ambitieux concernant la chasse. Notre commission a donc apporté des modifications substantielles au projet de loi, en visant quatre objectifs principaux. Nous avons tout d'abord souhaité améliorer la gouvernance du futur établissement public, afin de garantir une représentation plus équilibrée des différentes parties prenantes. Sensible à la place particulière qu'occupe le monde cynégétique dans les politiques en faveur de la biodiversité, la commission a renommé l'Office français de la biodiversité : « Office français de la biodiversité et de la chasse ». Elle a également modifié en profondeur son mode de gouvernance, dans le souci de lui assurer une représentativité et une efficacité renforcées. Ainsi, elle a supprimé la règle de la majorité acquise aux représentants de l'État, lui préférant un conseil d'administration moins pléthorique, mais rassembleur de toutes les parties concernées, dont certaines avaient été jusqu'alors oubliées. Dans un second temps, notre commission s'est montrée soucieuse d'étoffer les pouvoirs de police judiciaire dont sont attributaires les inspecteurs de l'environnement, et plus généralement les fonctionnaires et agents publics chargés d'une mission de police de l'environnement. Elle a, pour ce faire, retenu une approche équilibrée : favorable à un renforcement de leurs pouvoirs de coercition, sur lesquels le texte initial était presque muet, elle s'est toutefois refusée à leur conférer des pouvoirs calqués sur ceux des officiers de police judiciaire. Sans nier les difficultés auxquelles sont exposés les agents de police spéciale de l'environnement, il ne nous a pas semblé approprié de les doter de toutes les prérogatives d'officiers de police judiciaire, sans qu'ils aient préalablement reçu la reçu la formation nécessaire ou sans qu'ils disposent des locaux adéquats. La commission s'est donc attachée à étendre le périmètre de leurs pouvoirs de contrainte, tout en considérant que l'activité répressive devrait rester le dernier recours de cette police spécifique. Le troisième objectif visé par notre commission a été d'enrichir les dispositions du texte relatives à la chasse. Toutes les chasses doivent être prises en compte dans leur diversité. Dans nombre de territoires, la chasse reste une activité populaire, accessible à un large public, aussi bien à des jeunes ouvriers ou artisans qu'à des retraités aux revenus modestes. Ainsi, compte tenu de leur rôle incontournable dans nos territoires, nous avons notamment conforté les missions des fédérations départementales en matière de gestion du patrimoine naturel et d'organisation des activités de chasse.

d'apporter 10 euros par permis validé aux fédérations des chasseurs, en complément de l'obligation incombant à chacune d'entre elles de dépenser au moins 5 euros par permis en faveur de la protection de la biodiversité. Chaque fédération départementale recevra directement cette contribution à due concurrence du nombre de ses adhérents, tandis que la Fédération nationale des chasseurs sera chargée de gérer un fonds permettant d'assurer une péréquation complémentaire entre fédérations locales.

la lutte contre les dégâts de grand gibier, qui constituent un véritable fléau dans certains territoires, en particulier pour les agriculteurs et les forestiers. À cette fin, nous avons accru les pouvoirs du préfet en matière de plans de chasse en cas d'augmentation des dégâts dans un département. Notre commission a par ailleurs décidé de mesurer avec certains critères le nourrissage des sangliers, ainsi que la vente et le transport de ces animaux, pour mieux maîtriser les populations et les risques sanitaires, lesquels sont d'actualité. En matière de gestion adaptative, la commission a tenu à ce que le nouveau dispositif ne se traduise pas par des contraintes excessives pour les chasseurs, notamment en atténuant les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation de transmettre les données de prélèvement. ailleurs, nous avons complété le projet de loi par plusieurs dispositions visant à améliorer la protection du patrimoine naturel. Outre l'introduction dans le code de l'environnement d'une définition de la géodiversité, nous avons élargi le périmètre des aires marines protégées et clarifié les critères de reconnaissance des zones humides. Enfin, la sécurité liée à la pratique de la chasse doit être améliorée, notamment dans la visibilité des chasseurs. Renforcer les mesures de sécurité sera bénéfique à tous, et en premier lieu aux chasseurs eux-mêmes. Au total, le texte adopté par notre commission présente un projet de réforme plus équilibré, qui permet de donner toute sa place aux différentes parties prenantes. À ce titre, nous nous réjouissons que ce projet de fusion se présente dans une atmosphère constructive et apaisée. Chacun a compris qu'il était indispensable de sortir d'une opposition stérile et caricaturale entre de supposés défenseurs et de supposés opposants de la biodiversité. Il est nécessaire d'agir en privilégiant des solutions partagées, concrètes et pragmatiques, élaborées au plus près du terrain. C'est ainsi que nous assurerons une meilleure protection de la biodiversité. Je conclurai mon propos par la question du financement du futur établissement public, qui suscite les plus vives inquiétudes de notre commission. En effet, à l'issue de la loi de finances pour 2019 et de plusieurs arbitrages complémentaires, le budget de l'établissement sera confronté à près de 40 millions d'euros

Les débats que nous aurons, ensemble, permettront, je l'espère, de clarifier ces incertitudes financières. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, souvent décriés, les chasseurs sont pourtant des acteursincontournables de la biodiversité. Fins observateurs de lanature, ce sont les premiers à constater les évolutions de notreenvironnement. Je ne puis que regretter que leur rôle ne soit pas reconnu à sajuste valeur. Les chasseurs n'ont en effet pas attendu ce projetde loi pour conduire des actions en matière de biodiversité, et les montants engagés dépassent bien souvent les 5 euros par permis de chasser. Le Gouvernement propose de leur transférer deux compétences : la gestion des plans de chasse et celle des ACCA, ce dont je me félicite. Le rôle des ACCA n'est plus à démontrer, chacun en conviendra. Il faut cependant veiller au maintien de ces associations qui contribuent à la régulation du gibier et de la biodiversité en favorisant le regroupement de terrains morcelés de petite taille. Elles sont la garantie d'une chasse populaire.

Comme vous, madame la secrétaire d'État, nous pensons que la dénomination d'un établissement est importante, qu'elle renvoie à son identité et à ses ambitions. Au regard de leur rôle en matière de biodiversité, nous avons estimé que les chasseurs devaient avoir toute leur place au sein de ce nouvel établissement. C'est pourquoi nous l'avons rebaptisé « Office français de la biodiversité et de la chasse ». Nous avons également cherché à rééquilibrer son conseil d'administration en faveur des chasseurs, mais aussi de deux autres acteurs importants, dont le coeur de l'activité est lié à la nature. Je veux bien entendu parler des agriculteurs et des forestiers. Sur un sujet aussi important que la biodiversité, l'État doit savoir convaincre ses partenaires et rechercher le consensus. L'État n'a la majorité ni dans Parcs nationaux de France ni à l'ONCFS. Ces établissements n'en sont pas moins bien gérés. Il n'y a donc aucune raison que ce soit différent pour l'OFB. C'est pourquoi nous avons proposé que l'État n'ait pas la majorité, mais uniquement un droit de veto. Tel est le sens des amendements que j'ai portés, et qui ont été adoptés par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Pis, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous : il manque 41 millions d'euros dans le budget du nouvel établissement. Les agences de l'eau participeront au financement hauteur de 258 millions d'euros. Elles devront en outre financer la promesse de l'État de mettre 10 euros pour 5 euros versés par les chasseurs, soit 11 des 41 millions manquants. Une présence de l'État dans le financement de l'OFB à hauteur de 30 millions, on aimerait y croire, mais nous connaissons tous Bercy ... Je crains que les agences de l'eau ne soient de nouveau mises à contribution, et ce aux dépens des communes et des EPCI. Ces prélèvements sur les agences de l'eau sont intolérables. Ils sont contraires aux directives européennes relatives à l'eau et au principe selon lequel l'eau doit payer l'eau. Comment les agences pourront-elles, demain, réaliser leurs investissements en matière d'eau potable et d'assainissement, si nous continuons à les ponctionner de la sorte ? Présenter des réformes non ficelées sur le plan budgétaire, cela devient une manie, une très mauvaise habitude. En nous renvoyant au prochain projet de loi de finances, vous desservez, madame la secrétaire d'État, la réforme que vous proposez, et vous desservez la biodiversité que vous entendez défendre. Comme Jean-Claude Luche et Jean-Noël Cardoux, avec lesquels j'ai travaillé en bonne intelligence, et nos collègues sénateurs, nous serons au rendez-vous des débats budgétaires pour réexaminer le circuit de financement du nouvel établissement et revoir la contribution des agences de l'eau. En conclusion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi sous réserve des amendements qu'elle a adoptés et des réponses apportées aux interrogations que soulève une réforme dont la soutenabilité financière n'est pas assurée. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, « si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterai quand même un pommier Je reprends cette phrase de Martin Luther King à mon compte, tant il est primordial dans la lutte pour la préservation de la biodiversité de ne jamais baisser les bras. Mon engagement est ancien dans ce combat. Il m'a mené sur de nombreux chemins, un peu partout dans le monde, à la rencontre de multiples institutions, organismes et personnes concernés. Je puis vous confirmer qu'il existe de très belles initiatives, dans tous nos territoires métropolitains et ultramarins : chaque action, même la plus anodine, compte, et contribue à ce combat. Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, enrayer l'effondrement de la biodiversité est plus que jamais capital. Le maintien de la biodiversité est une condition de notre propre survie ; nous en sommes un des éléments essentiels. La biodiversité est tout à la fois le tissu vivant de notre planète et notre pharmacie elle fournit en biens et services près de deux fois la valeur de ce que produisent les humains chaque année ; plus de 70 % des cultures que nous consommons dépendent d'une pollinisation animale.

compte tenu du rythme actuel de leur disparition, cent à mille fois supérieur au taux naturel d'extinction. La crise d'extinction actuelle est bien plus rapide, et elle est quasi exclusivement liée aux activités humaines. humaines. Avec ses outre-mer, la France se situe parmi les dix pays abritant le plus grand nombre d'espèces mondialement menacées. Les milieux naturels sont fragilisés ou détruits par les activités humaines : sur l'ensemble de la planète, 60 % d'entre eux

perd ses espaces cultivables. J'ai récemment remis un rapport au Premier ministre sur les « zones humides ». Le constat est sans appel : ces terres d'eau, milieux dont les bienfaits sont inestimables pour l'homme, continuent de disparaître à un rythme accéléré. Heureusement, le thème de la biodiversité et de sa préservation s'impose de plus en plus dans les débats publics ; les jeunes générations, à l'image de la Suédoise Greta Thunberg, sont de plus en plus réceptives à l'idée d'interroger notre place, notre rôle au sein de la biodiversité et l'impact de nos activités, en lien avec la problématique du changement climatique.

Les pays membres de l'ONU, les pays européens et l'Union européenne ès qualités se sont lancés dans cette formidable aventure dont le succès conditionne la réussite de l'accord de Paris. Le plan Biodiversité lancé en 2018 répond en partie à cet Il faut aussi des opérateurs publics puissants et efficaces. La gouvernance est en effet un enjeu majeur de la préservation et de la gestion de la biodiversité. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires et moi-même nous félicitons donc de la création de l'Office français de la biodiversité, qui sera, nous en sommes certains, un opérateur clé pour restaurer et protéger la biodiversité de façon efficace. À l'Assemblée nationale, j'avais été le promoteur législatif de l'Agence des aires marines protégées

des rapporteurs -humains et financiers : je partage à cet égard les inquiétudes exprimées sur les 40 millions d'euros manquants. L'office doit être doté des moyens d'agir. Le projet de loi semble à première vue assez technique, mais il traduit en réalité un portage politique affirmé pour répondre aux enjeux de la biodiversité en France. Ce nouvel office devrait permettre d'accroître l'efficacité des politiques de l'eau et de la biodiversité par une meilleure connaissance, surveillance, préservation et gestion des espèces et milieux. Le renforcement de la police de l'environnement sur le terrain, au plus près des besoins, et l'adossement à une expertise scientifique et technique reconnue étaient bien sûr indispensables. le travail du rapporteur Jean-Claude Luche et de la rapporteure pour avis Anne Chain-Larché pour les améliorations déjà apportées à ce projet de loi par notre assemblée en commission. Le travail en bonne intelligence avec toutes les parties intéressées- chasseurs, agriculteurs, acteurs économiques, organismes privés et publics, ONG, scientifiques -sera également primordial pour le bon fonctionnement de ce nouvel office.

de faire une chose, on la manque. » Ce moment est aujourd'hui arrivé. Chaque pierre sera utile pour fortifier l'édifice de la préservation et de la reconquête de la biodiversité. Espérons que ce nouvel office sera l'une de ces pierres ! La parole est

débats. Ce texte est celui des engagements tenus, par le chef de l'État et le Gouvernement, par le monde de la chasse, mais aussi par les environnementalistes. C'est le texte de tous les acteurs de la protection des écosystèmes. À ce titre, il mérite d'être salué. Voté à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale, le présent projet de loi va permettre d'envisager des pratiques plus rationnelles et une meilleure protection de l'environnement. C'est un projet de loi à la fois ambitieux, courageux et visionnaire ; il est équilibré à l'égard de l'ensemble des partenaires du monde rural. Il s'inscrit dans un pari audacieux, auquel j'adhère totalement, car il s'agit d'assurer et d'assumer le développement de la chasse française dans tous nos territoires ruraux. Il s'agit également de porter l'idée que la chasse doit s'adapter, se moderniser, s'ouvrir pour gérer plus efficacement la faune sauvage, responsabiliser les gestionnaires des territoires, partir à la reconquête de l'opinion publique et promouvoir une chasse durable.

Chacun veut la survie des différentes espèces, et personne ne souhaite mettre à mal les espèces menacées. La gestion adaptative doit s'appliquer seulement aux espèces qui posent des problèmes,

J'ai l'intime conviction que la réforme sera totalement financée et que l'État assumera ses choix. Mais comme beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, je pense que les flux croisés qui sont indispensables pour cette première saison doivent faire l'objet d'une renégociation rapide pour la prochaine loi de finances. Pour être très clair, j'ai toujours j'ai toujours pensé que l'argent de la chasse devait payer la chasse, que l'argent de l'eau devait d'abord payer l'eau et que les missions régaliennes de police rurale et d'expertise sur la biodiversité terrestre devaient être prises en charge de l'État. En conclusion, mes chers collègues, que des esprits chagrins pensent encore que le Président de la République et le Gouvernement ne savent pas négocier les réformes avec les corps intermédiaires, notamment ruraux, nous avons la démonstration du contraire avec ce projet de loi qui a été bien négocié.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'idée de rassembler au sein d'un opérateur unique l'ensemble des opérateurs de la biodiversité n'est pas nouvelle. elle avait émergé, il y a déjà quelques années, avec le Grenelle de l'environnement. Ce n'est pas un hasard si le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. En effet, de par leurs missions respectives, l'AFB et l'ONCFS sont complémentaires, et leur fusion permettra l'émergence d'un opérateur public cohérent et puissant, présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Cette fusion marque, en outre, un changement d'approche et la volonté affirmée de ne plus séparer gestion de la biodiversité et activités cynégétiques. En effet, l'AFB a vocation à appuyer les services de l'État dans la gestion des espaces naturels et la police de l'eau. Elle organise la connaissance en matière de biodiversité, elle fournit aux acteurs locaux les données et l'expertise dont ils ont besoin. L'ONCFS, quant à lui, fait partie intégrante de la politique de préservation de la biodiversité, ne serait-ce que par ses activités « non cynégétiques » de connaissance et d'expertise, de police de l'environnement, de lutte contre le trafic d'espèces menacées, ou encore de suivi des espèces protégées comme le loup. Dès lors, comment ne pas souscrire à l'objectif de rassembler et de renforcer les prérogatives des inspecteurs de l'environnement des deux opérateurs en un service unique, afin de permettre une action mieux coordonnée et mieux répartie sur le territoire Notons cependant que, après l'Agence nationale de la cohésion des territoires, après la loi d'orientation des mobilités, ce gouvernement est devenu spécialiste en « plomberie administrative Regrouper des services, des administrations pour tenter d'améliorer les politiques publiques peut être utile et louable, mais tout bon plombier sait que la réparation de fuite, le colmatage, ne remplacera jamais un réseau régulièrement entretenu. En d'autres mots, on ne fait pas d'action publique de long terme sans moyens financiers. Ainsi, alors que nous n'avons pas vu dans le dernier projet de loi de finances la couleur des 600 millions d'euros supplémentaires promis pour le plan Biodiversité, ce nouvel office est créé avec près de 40 millions d'euros annuels non financés. L'État s'est purement est simplement désengagé progressivement du financement de l'AFB et de l'ONCFS, remplaçant ses contributions et subventions par des ponctions sur les agences de l'eau, comme cela a été rappelé. En plomberie, nous appelons cela du siphonnage ! Cette contribution des agences de l'eau est comprise entre 240 millions d'euros et 260 millions d'euros pour l'Agence française pour la biodiversité et entre 30 et 37 millions d'euros pour l'ONCFS.

La seule fiscalité de l'eau, assise sur les redevances aux agences de l'eau, ne peut financer l'ensemble de la biodiversité. En revenant sur le principe selon lequel « l'eau paye l'eau », admis par l'ensemble de nos concitoyens, vous prenez le risque, une nouvelle fois, de créer de l'incompréhension. Nous sommes passés de « l'eau paye l'eau », à « l'eau paye l'eau et la biodiversité » et maintenant à « l'eau paye l'eau, la biodiversité et la chasse ». Ponctionner les agences, c'est limiter les investissements en matière d'eau potable et d'assainissement, donc agir moins pour la biodiversité. un comble, alors même que les Assises de l'eau ont mis en lumière d'importants besoins liés aux conséquences des changements climatiques sur l'état et la répartition des masses d'eau ! Encore une fois, si la question du financement est la principale faiblesse de ce texte, celui-ci fait naître une autre inquiétude, qui lui est directement liée : le déploiement de l'office dans les territoires. Comme l'a souligné la rapporteure à l'Assemblée nationale, dans de nombreux départements, les effectifs planchers de l'office ne sont pas atteints ... La présence des agents sur le terrain est pourtant la raison d'être d'une telle administration, qui ne pourra pas préserver la biodiversité depuis des bureaux parisiens. Néanmoins, vous nous avez confirmé en commission une baisse continue de 2 % des effectifs. Je ne prendrai qu'un exemple qui me tient à coeur : celui de la « brigade loup ». Ses 11 agents, qui ont fait montre de toute leur efficacité, ont vu leurs CDD non renouvelés avant d'être prolongés, au bout d'un long suspense, des contrats d'avenir Cette situation précaire n'est pas acceptable, tout d'abord pour ces agents et leurs familles, mais aussi au regard de la transmission de l'expérience qu'ils ont acquise, indispensable pour favoriser la cohabitation entre le prédateur et les activités d'élevage, alors que la population de loups est en croissance exponentielle. Au-delà de ces deux écueils importants, l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale a permis de bâtir un bon compromis, dont je me félicite. Ce texte équilibré a permis de trouver un consensus entre les chasseurs et les associations de protection de l'environnement. Ce compromis, cet équilibre fragile, a malheureusement été mis à mal lors de l'examen du texte ici en commission. Je le regrette, dans l'intérêt des activités cynégétiques et pour la préservation de la biodiversité.

La transformation du nom de l'Office français de la biodiversité en Office de la biodiversité et de la chasse est assez symptomatique : cela revient à nier une reconnaissance pourtant si souvent souhaitée.

Nous tenterons, avec nos amendements, lors du débat, de retrouver le compromis de l'Assemblée nationale et de revenir à un texte plus équilibré. Il faut sortir des postures caricaturales, comme le soulignait M. le rapporteur. Alors que notre planète connaît sa sixième extinction de masse, laquelle est directement liée aux activités humaines, j'espère que le Sénat, chambre des territoires, gardera raison et saura défendre notre patrimoine commun, la diversité de la vie. La

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout le monde a conscience désormais du fait que la biodiversité fait partie du patrimoine commun de l'humanité, que sa préservation est essentielle, qu'elle est pour nous un devoir. En effet, nous avons pris acte que la biodiversité était menacée. On peut le souligner, il n'y a pas de « biodiversito-sceptiques Cela a déjà été mentionné, la France héberge quelque 10 % de la biodiversité de notre planète, dont 90 % dans les territoires ultramarins. C'est dire la richesse de la nature outre-mer Pourtant, le constat de la disparition des espèces s'impose à tous. La communauté scientifique est unanime sur la gravité et l'urgence de la situation. La moitié des espèces vivantes pourrait disparaître d'ici à un siècle, compte tenu du rythme d'extinction des espèces animales. Cette dégradation de la biodiversité et son rythme effréné trouvent très essentiellement leur origine dans les activités humaines : réduction et fragmentation des espaces naturels, déforestation, pollution de l'eau, des sols et de l'air, changement climatique, surexploitation des ressources, trafic d'espèces, etc. Il convient donc de nous doter des structures les plus adaptées, cohérentes et efficaces pour agir en la matière. L'Agence française pour la biodiversité, née de la loi du 8 août 2016, avait déjà regroupé plusieurs établissements publics, comme cela a déjà été indiqué. L'intégration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'Agence française pour la biodiversité avait été envisagée lors les réflexions relatives à la création de Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a donc pour objet de fusionner ces deux établissements sous l'égide d'un Office français de la biodiversité et de la chasse, ainsi que la commission vient de le renommer, et qui verra le jour le 1 janvier prochain. La fusion de ces deux établissements, qui est d'ailleurs souhaitée par la majorité des acteurs de la biodiversité, nous apparaît cohérente. Elle s'inscrit dans la continuité de la Stratégie nationale pour la biodiversité. Elle conforte l'idée d'une culture commune, rapproche les expertises complémentaires de ces établissements, et renforce l'action territoriale, ainsi que la police de l'environnement. Je tiens à souligner le travail de précision des missions du futur office auquel a procédé l'Assemblée nationale et l'esprit de concertation dans lequel l'examen du texte en commission s'est déroulé, permettant l'adoption d'avancées telles que le renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l'environnement, ou encore l'inscription dans la loi de la contribution de 10 euros de l'État par permis de chasser. chasser. Concernant la chasse, soulignons certaines dispositions de ce projet de loi, notamment le renforcement de la sécurité qu'il opère, l'amélioration de l'indemnisation des dégâts de gibier ou encore la gestion adaptative des espèces. Cependant, nous resterons particulièrement vigilants sur certains points. Comme vous le savez, madame la secrétaire d'État, la question du financement de ce nouvel office fusionné reste bien trop incertaine à nos yeux. Avec la baisse du prix du permis de chasser national, les charges supplémentaires correspondant aux nouvelles missions transférées, et l'abondement de l'État de 10 euros par adhérent ayant un permis de chasser validé dans l'année, ce sont 40 millions d'euros de financement pour 2020 qui restent en suspens. Concernant l'organisation de l'office, nous souhaiterions aussi être assurés que cette fusion ne se résumera pas à un moyen de faire des économies sous prétexte de mutualisation.

chez eux un sentiment d'instabilité dont nous devons être conscients. Enfin, nous sommes convaincus qu'il existe entre le monde de la chasse et la protection de la nature une convergence des objectifs et une complémentarité justifiant la fusion de ces deux établissements. Nous devons donc garder à l'esprit que cela ne tombe pas sous le signe de l'évidence pour tous. Nous espérons que cet office pourra être un outil pertinent et efficace de lutte contre le déclin de la vie sauvage. La

Dantec. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, monsieur le président de la commission, je me permets de commencer cette intervention par une exclamation de surprise : déjà ! Cette fusion, au sein d'un même office, des acteurs de la biodiversité et de la chasse semblait en effet encore totalement inaccessible il y a moins de trois ans, au moment de la discussion de la loi pour la reconquête de la biodiversité, Nous étions pourtant déjà un certain nombre à considérer que ce regroupement des acteurs de la nature, et notamment des agents exerçant une fonction de police de l'environnement, était nécessaire à une véritable politique de protection de la nature, qu'elle allait dans le sens de l'histoire. On nous répondait que les choses n'étaient pas mûres, que les différences, les méfiances ataviques, le fossé culturel entre les acteurs étaient bien trop importants pour permettre ce rassemblement, et qu'il fallait donc laisser du temps au temps. Nous ne pouvons donc que féliciter le Gouvernement et le Président de la République d'avoir réussi cette prouesse : avoir trouvé les arguments pour amener les uns et les autres à cette fusion. La création de l'office, avec dorénavant 2 700 agents publics équivalents temps plein travaillés, dote les politiques de biodiversité d'un outil important.

cette rapidité de la fusion entre l'AFB et l'ONCFS suscite, vous le savez, beaucoup de questions et d'inquiétudes des deux côtés. « Quelle est la véritable nature du entre entre l'État et les chasseurs ? », s'alarment les associations de protection de la nature. « La chasse ne sera-t-elle pas la perdante à terme de cette intégration, synonyme de perte d'influence ? », s'inquiètent les fédérations. Nous n'avons pas à ce stade, disons-le, la totalité de la réponse à ces questions. Mais il y a un pari, que j'assume avec beaucoup d'autres ici : celui que les intérêts communs des chasseurs et des non-chasseurs, unis dans la défense de notre patrimoine naturel et du fonctionnement des écosystèmes, sans lesquels il n'y a ni gibier ni espèces protégées, espèces protégées, deviennent plus importants que les seuls débats sur les dates d'ouverture et le niveau des prélèvements autorisés. Il y aura encore des confrontations, évidemment, mais espérons que cette culture commune s'imposera progressivement. Le Sénat en a d'ailleurs souvent donné l'exemple, et, sans vouloir mettre Jean-Noël Cardoux en difficulté, tant ces interventions seront scrutées par ses camarades, je voulais rappeler sur la loi relative à la biodiversité, il nous est arrivé, à lui et à moi, de défendre les mêmes amendements- le rapporteur de l'époque, Jérôme Bignon, que je salue tout particulièrement pour son investissement sur ces enjeux, pourra en témoigner. Je soutiens donc le rapporteur dans sa volonté d'élargir la gouvernance de l'office, car il faut que tout le monde échange et discute, et je ne doute pas de la capacité de l'État à équilibrer soigneusement les représentations.

Il ne serait pas raisonnable de sortir la liste des espèces chassables issue de la directive Oiseaux de 2009 ; surtout, il va falloir arrêter de chasser les espèces en forte régression,

quand ces chasses seront de nouveau autorisées, grâce à une politique ambitieuse, portée ensemble par les chasseurs et par les écologistes, pour la préservation des biotopes et la lutte contre les pollutions, notamment chimiques est le sens, semble-t-il, d'une gestion adaptative des espèces et d'une chasse durable. Cela rejoint aussi les propos du ministre d'État François de Rugy : « Si une espèce voit son effectif augmenter, elle peut être chassée, et inversement. » Tout est dans le « et inversement » ... À propos de gestion adaptative des espèces, notre souci commun est quand même la démographie des chasseurs eux-mêmes. Plus de 2,2 millions de chasseurs en 1975, moins de 1,2 million en 2018,

Si je puis me permettre ce modeste conseil, le monde de la chasse, plutôt que de nourrir et d'élever quelques lobbyistes à l'action discutable, investir dans une communication nouvelle, sans s'engluer dans la défense de pratiques anciennes, condamnées à disparaître. Je voudrais vraiment vous convaincre que ces images d'oiseaux aux plumes collées et autres scènes contribuent à détourner les jeunes de cette activité, considérée comme d'un autre temps- pour ne pas employer de termes plus polémiques. Pour assurer son avenir, la chasse doit montrer son action bénéfique et souligner, avec l'appui de scientifiques et de données fiables, son impact positif sur l'évolution des espèces. Elle susciterait ainsi de nouvelles adhésions,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité s'inscrit dans un contexte de menaces et de pressions sans précédent pour la biodiversité. Ces pressions se traduisent dans tous les espaces naturels, agricoles et forestiers. Elles sont le fait de multiples phénomènes qui se conjuguent : changements climatiques, facteurs humains liés à la fréquentation grandissante, mais aussi fiscalité française sur le foncier défavorable aux espaces naturels et prolifération de gibiers. La Fédération nationale des chasseurs a pris une part importante dans les débats préalables à ce projet de loi. De ce fait, les chasseurs constituent la pierre d'angle du dispositif prévu dans le cadre de ce nouvel office. sont bel et bien essentiels à la régulation des populations de gibiers, et donc au maintien d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique, il convient que, dans un souci de légitimité et d'efficacité de l'institution, le projet de loi dont nous allons débattre appréhende le sujet de la biodiversité dans sa globalité, en posant les fondements d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs et d'une gestion partagée et équilibrée des espaces naturels, où chasseurs, agriculteurs, forestiers et usagers prendront en compte les réalités des uns et des autres. C'est aujourd'hui indéniable, l'agriculture comme la sylviculture sont les victimes des dégâts de gibier, devenus insoutenables. Pour la saison de 2017, les chasseurs français ont versé plus de 37 millions d'euros aux agriculteurs, et le coût global atteindrait près de 60 millions d'euros en 2018. C'est dire le poids financier supporté par les chasseurs, mais aussi l'évolution et l'impact négatif des déséquilibres cynégétiques sur des exploitations agricoles parfois en survie. la forêt, il n'existe pas de chiffres, car, puisqu'il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas d'inventaire. Néanmoins, sur le terrain, les dégâts de gibier intégralement assumés par les forestiers sont considérables et augmentent. Ils fragilisent une forêt déjà assaillie par les attaques de parasites, déstabilisée par les changements climatiques et par les déficits hydriques récurrents, et vulnérable aux incendies. une forêt dont les services écosystémiques en matière de biodiversité et de captation de carbone sont insuffisamment reconnus et soutenus, alors même que l'État et l'Europe envisagent zéro émission nette de carbone d'ici à Comme l'agriculture, cette forêt, gérée jusqu'à présent dans une logique multifonctionnelle, préservant la biodiversité et créatrice d'emplois, doit pouvoir s'appuyer sur des politiques publiques cohérentes. Pour cela, il est essentiel que ce projet de loi accorde une place légitime à l'ensemble des acteurs de ces espaces naturels, et prenne en considération, à trois échelons, les réalités de la filière forêt et bois : dans la gouvernance- en accordant une meilleure représentativité aux forestiers et en assurant la cohérence entre plan de chasse et plan d'aménagement forestier, qu'il soit public ou privé -, dans le cadrage juridique- en réaffirmant la pertinence du code forestier, de la procédure pénale forestière, et en confiant des prérogatives ajustées aux inspecteurs de l'environnement, notamment pour lutter contre les dépôts sauvages en forêt enfin, dans les orientations politiques- en se fondant sur le cadrage national décliné notamment dans les plans régionaux de la forêt et du bois et dans les commissions sylvo-cynégétiques, et en préservant le droit d'arbitrage du préfet. Autant d'éléments d'équilibres essentiels, qui figurent, pour la plupart, dans l'excellent rapport de notre collègue Jean-Noël Cardoux, et que je vous proposerai d'intégrer au texte présenté aujourd'hui. Nous souhaitons tous, mes chers collègues, parvenir à un compromis qui fera sens sur le terrain

plutôt qu'une tentative de marginalisation, la reconnaissance explicite que la chasse est un élément incontournable de la biodiversité, ce que nous avions déjà affirmé lors de la discussion de la loi de 2016.

alors que le monde de la chasse apportera à lui seul 45 millions d'euros au budget général de l'organisme. Troisième interrogation, la technicité et l'excellence de l'ONCFS, en matière d'études et de contribution à la biodiversité, seront-elles sauvegardées ?

beaucoup combattu pour cette direction unique lors de la discussion de la loi sur la biodiversité -permettra-t-elle de réprimer le grand braconnage et l'exploitation mercantile des espèces animales et végétales ?

Le comité des experts, qui est en place depuis quelque temps et qui va devoir statuer sur le contenu des espèces soumises à la gestion adaptative, sera-t-il suffisamment impartial et, surtout, utilisera-t-il le relais des associations spécialisées les chasseurs de gibier d'eau, de bécasses, de bécassines, ceux qui se consacrent journellement aux études, aux comptages, aux prélèvements d'ailes -afin de déterminer des sexe-ratios et des âge-ratios crédibles ? C'est la technique de pointe de gestion adaptative appliquée aux États-Unis et au Canada,

permettra-t-il d'attirer de nouveaux chasseurs- c'est son objectif -, qui pourront ainsi découvrir de nouveaux modes de chasse sur l'ensemble du territoire ? Au sujet des dégâts de grand gibier- un dialogue apaisé pourra-t-il s'établir entre les acteurs du monde rural que sont les agriculteurs, les chasseurs et les forestiers, avec comme toile de fond la menace de la peste porcine africaine ?

que le coup de sifflet final ne soit donné par la peste porcine africaine, qui pourrait envahir l'ensemble du territoire français, avec les catastrophes économiques que cela pourrait engendrer. la taxe à l'hectare, qui est au coeur du problème, y compris sur les territoires non chassés, sera-t-elle suffisante pour faire face à cette charge ? Sera-t-elle supportable pour les petites fédérations ? J'ai introduit dans mon amendement à ce sujet un élément amortisseur pour établir un rapport entre la surface des territoires chassables et le nombre de chasseurs. Nous sommes là au coeur du débat, je suis encore en contact avec la Fédération nationale des chasseurs pour tenter

permettra-t-elle d'enrayer l'idéologie végane et antispéciste, ultra-minoritaire et irréaliste, ayant l'oreille complaisante des médias ?

j'y reviendrai lors de la discussion de l'amendement. Il faut le savoir, dans certaines régions, en particulier dans les régions de tradition de chasse de grand gibier, comme l'est de la France, les installations fixes- miradors ou échelles de chasse -qu'utilisent les chasseurs sont

Je ne reviendrai pas sur les sujets dont le Sénat a déjà beaucoup débattu- fermeture des commerces, mobilité, désertification médicale, absence de supports de communication -, vous

si l'Office français de la biodiversité n'a pas vu le jour dès 2016, au moment de la création de l'Agence française pour la biodiversité, c'est que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale de la chasse n'avaient alors pas assez de visibilité sur l'avenir de ce nouvel établissement. Aujourd'hui, il semble que tout soit réuni pour réussir cette union. La lutte pour la sauvegarde de la biodiversité sur notre territoire métropolitain et ultramarin est au coeur des missions des deux organismes. La mise en commun de leurs compétences et leurs sensibilités complémentaires seront des atouts essentiels. Avec la création de cet office, la répartition des équipes sur le terrain sera plus homogène, l'ONCFS ayant des effectifs plus importants déployés dans les départements. Les pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement seront renforcés. Cette compétence, qui répond aux nécessités constatées sur le terrain, permettra de rendre la police de l'environnement plus efficace et plus rapide. Concernant les fédérations de chasseurs, le financement de 5 euros par permis de chasse pour la protection de la biodiversité me paraît justifié, mais inscrivons dans la loi que l'État apporte une contribution équivalant au double

deux mètres de haut autour de vastes propriétés de plus de mille hectares. Ces grillages sont non seulement une catastrophe visuelle, mais encore une aberration pour la mobilité des grands animaux et pour la préservation de la biodiversité.

mais il sera toujours possible de clore une parcelle pour sa régénération ou pour une nouvelle plantation. La gestion adaptative, fondée sur la communication des prélèvements de certaines espèces, en lien étroit entre les scientifiques et la Fédération nationale des chasseurs, permettra une meilleure gestion de la biodiversité. Le décret listant les espèces ouvertes à la chasse pourrait également être revu, à terme, pour y intégrer certains spécimens qui, par leur nombre, causent des nuisances et sont susceptibles de perturber les écosystèmes. Je pense en particulier on en compte des milliers sur la Loire, qui vont piller les étangs de Sologne, au grand désarroi des pisciculteurs. Ce nouvel office de la biodiversité n'a pour l'instant pas de financement bien lisible. En l'état actuel, il semblerait qu'il manque encore environ 40 millions d'euros dans le budget, et ce ne sont pas les agences de l'eau, grandes contributrices au financement de l'ONCFS, qui devront supporter cette différence.

J'ajoute qu'il est positif que la chasse et la pêche soient intégrées à cette politique et qu'elles participent à la régulation et à la préservation des écosystèmes dans notre pays. La parole est à M. Michel Magras.

la logique de rationalisation qui préside au projet de création de l'Office français de la biodiversité ne doit pas conduire à sacrifier l'attention particulière que méritent les outre-mer en cette matière, et que l'organisation de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, a reflétée jusqu'ici de manière remarquable. Le législateur de 2016, sans doute soucieux de sanctuariser cette place, avait inscrit dans la loi la création d'un « comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer

Madame la rapporteure, chère collègue, permettez que je m'associe à l'expression de vos regrets pour déplorer à mon tour que le Gouvernement n'ait pas concédé aux outre-mer leur juste place dans l'architecture du nouvel établissement, eu égard à la richesse, à l'ampleur et à la complexité de la biodiversité ultramarine. Le rappel de quelques chiffres me semble opportun, même si nous finissons tous par les connaître

carrés de récifs et de lagons- la barrière récifale néocalédonienne est la deuxième au monde et celle de Mayotte est un exemple unique de double barrière -, et 8 millions d'hectares de forêt guyanaise, une des dernières forêts primaires au monde. ne constituent pourtant qu'une énumération brève, bien qu'emblématique, de l'extrême richesse patrimoniale française située outre-mer, où il est traditionnel de considérer que se trouve plus de 80 % de la biodiversité nationale.

La délégation aux outre-mer, que j'ai l'honneur de présider, est très attentive à ces deux aspects, qui font l'objet d'une association avec l'Agence française pour la biodiversité, sous la forme d'un cycle triennal de colloques, avec une déclinaison par grand bassin océanique, contribuant ainsi à accroître la vigilance et à assurer la visibilité du patrimoine écologique ultramarin. À ce titre, nous sommes les témoins, et les associés privilégiés, de l'immense travail accompli, du dynamisme et de l'implication de l'AFB pour la préservation et la valorisation de la biodiversité ultramarine.

En outre, si la délégation aux outre-mer saisit chaque occasion de rappeler la place de sentinelle des outre-mer, elle n'oublie pas que ces territoires sont aussi les premières victimes du dérèglement climatique, conférant ainsi à la France une responsabilité particulière.

à démontrer l'absolue nécessité d'une structure gardienne de la politique de préservation et de valorisation de la biodiversité ultramarine au sein du futur Office français de la biodiversité.

L'exemple de la chasse en Guyane, qui sera probablement évoqué dans nos débats, est une nouvelle illustration de la complexité ultramarine que j'évoquais. Cette pratique doit être appréhendée de manière à trouver l'équilibre entre l'encadrement et la préservation d'une activité de subsistance aux règles ancestrales. Dans cette optique, la réforme de la chasse guyanaise devra être conduite en concertation étroite avec les chasseurs, en gardant en mémoire qu'elle revêt une dimension de protection patrimoniale et de préservation de pratiques de subsistance pour les populations amérindiennes. J'en terminerai par quelques mots sur le renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l'environnement ; la collectivité de Saint-Barthélemy, compétente en matière d'environnement, sera certainement amenée à solliciter une extension, adaptée

comme l'a souligné notre collègue Jean-Michel Houllegatte à la fin de son intervention, l'un des sujets à mettre en exergue de ce texte est bien la recherche de convergence entre deux mondes que l'on oppose souvent. Si l'on veut caricaturer, il y a, d'un côté, les défenseurs de l'écologie, qui ont forcément raison, car leur cause est noble, contre, de l'autre, les chasseurs, qui ont forcément tort, car leur objectif est de tuer des animaux. Il est donc pour le moins audacieux de les réunir, et même de les amener à fusionner au sein d'une même structure ; c'est comme marier la carpe et le lapin Le souhait d'une grande partie de mes collègues est d'ajouter au nom de l'Office français de la biodiversité la mention « et de la chasse ». Cela ne me semble pas être indécent ; c'est même plutôt légitime, puisque cet office va naître de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité

Ce débat sur le nom pourrait n'être qu'un détail ; il est pourtant primordial. Il s'agit, en effet, d'un miroir de l'évolution de notre société, dans laquelle il est de bon ton de rester dans le « politiquement correct » et d'abonder dans le sens des réseaux d'influence. Or, contre cette réforme, ces réseaux sont nombreux. travers du seul prisme de certains lobbies, la chasse est évidemment à bannir ; son image est réduite à des monstres qui abattent les animaux. Pourtant, si l'on peut effectivement condamner ceux qui ont pour seule motivation le chiffre d'animaux abattus, on peut aussi, en étant honnêtes, considérer qu'il ne s'agit que d'une minorité de chasseurs. La grande majorité doit être vue comme un acteur important du maintien de la biodiversité. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, dont je suis élu, déclare : « Chasse et pêche participent à notre culture du partage, du vivre ensemble, du bien manger et du bien vivre qui est l'âme de cette région. Sentinelles de la nature, les chasseurs ont toute leur place dans les campagnes et nos montagnes, comme les pêcheurs dans les lacs et rivières. » On retrouve ce bain de nature avec Marcel Pagnol, qui relate, dans, les exploits de son paternel durant une partie de chasse dans les collines du massif du Garlaban. Dans nos territoires ruraux, la chasse est effectivement une culture, une tradition qui rend service à l'environnement. Chaque année, en France, les chasseurs entretiennent et plantent plus de 20 000 kilomètres de haies et bosquets, pérennisant ainsi les atouts de ces architectures naturelles. Des milliers de mares, naturelles ou créées par l'homme, parfois alimentées par des fossés ou des canaux, sont entretenues par les chasseurs, qui assurent ainsi leur préservation. Ces micro-milieux offrent un intérêt écologique incontournable. Les chasseurs ont également une action forte de régulation du gros gibier. La prolifération des cervidés et des sangliers cause d'énormes dégâts pour l'agriculture et les forêts. Dans l'Hérault, les indemnisations des dommages causés par les sangliers sont passées, en quelques années, de 120 000 euros à 360 000 euros

J'assistais, samedi dernier, à l'assemblée générale des chasseurs de l'Hérault. À la tribune, le président Jean-Pierre Gaillard avait invité des agriculteurs, des forestiers touchés par des dégâts importants dus au grand gibier, des élus de la métropole montpelliéraine, le vice-président des randonneurs de l'Hérault ... soit beaucoup de personnes qui sont souvent opposées. La volonté du président, partagée par tous, est de bâtir une stratégie pour cohabiter sur les mêmes territoires. C'est la solution : n'opposons pas les genres, mais construisons ensemble. Dans une société où il est plus facile de porter des jugements que de se comprendre, les chasseurs veulent qu'on leur reconnaisse le droit d'exister. Les chasseurs vont, certes, voir le tarif de leur permis national baisser,

C'est pourquoi, au même titre que pour les 5 euros, nous aimerions que cette contribution soit inscrite dans la loi. Que dire des 41 millions d'euros de financement manquants ? Comment allez-vous trouver les budgets ? Une nouvelle ponction sur les agences de l'eau sera-t-elle programmée ?

Je voudrais simplement vous dire mon optimisme. Je pense que l'équilibre dont il a été beaucoup question est à notre portée. Ce texte est en effet le résultat d'une grande concertation, comme l'ont souligné les sénateurs François Patriat, Jérôme Bignon, Ronan Dantec

qui s'est assez largement exprimé en dehors de cet hémicycle entre des parties prenantes que nous n'avons pas besoin d'opposer, sans échange de gros mots, ni d'un côté ni de l'autre, peut également être atteint au sein de cet hémicycle.

On y retrouve de nombreuses références relatives aux milieux aquatiques et à la gestion de l'eau. Il s'agit de savoir, en pratique, comment vont s'articuler les missions de l'OFB et celles des agences territoriales de bassin. Les missions des fonctionnaires en charge de ces politiques vont-elles se télescoper ? Je suis bien consciente que l'Agence française de la biodiversité, jeune ancêtre de l'OFB,

ailleurs, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a substantiellement étoffé les missions du nouvel établissement. Elle a également précisé les contours de la mission relative aux politiques de l'eau et de la biodiversité en réaffirmant leur ancrage à l'échelon territorial et en déclinant leurs diverses composantes, au 4° de l'alinéa 12. Cette réaffirmation de l'ancrage territorial des missions interpelle véritablement les acteurs de terrain. Pouvez-vous préciser vos intentions ? En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de l'OFB, vous avez déclaré en commission souhaiter que son financement soit budgétaire et ne sollicite pas les agences de l'eau. Toutefois, les arbitrages n'étant pas rendus, vous n'êtes pas allée plus loin à ce stade. Quand on voit qu'il manque déjà 40 millions d'euros pour financer ce nouvel office et que les budgets des agences de l'eau sont continuellement ponctionnés, c'est inquiétant. Et cela soulève surtout une question simple : quelle est la volonté du Gouvernement sur la pérennité des agences de l'eau ?

dans le cadre de conventions, mener des actions dans les collectivités d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna. De quelle manière ces conventions pourront-elles être concrètement mises en oeuvre

Par ailleurs, la France a pris, dans le cadre du, une initiative remarquée pour l'adaptation, la biodiversité et la résilience dans le Pacifique. De nouveaux projets ou de nouveaux financements sont-ils à l'ordre du jour au titre de cette initiative ? Les collectivités françaises, éminemment concernées, seront-elles éligibles à ces projets comme le seront les États insulaires du Pacifique ? Enfin, où en sommes-nous de l'« équivalent fonds vert » pour les outre-mer du Pacifique ? Notre biodiversité, dans le Pacifique, est formidablement riche. Elle est aussi incroyablement fragile et nécessite d'être protégée.

l'effondrement massif de la biodiversité sur terre est une réalité malheureusement de plus en plus visible pour chacun d'entre nous : moins d'oiseaux moins d'insectes, moins de vers de terre ... Or la biodiversité, c'est la vie, tout simplement. La biodiversité, c'est un vaste tissu d'interactions constantes entre les espèces, nous compris. Sans le maintien de la biodiversité, nous pourrions être confrontés à une crise alimentaire mondiale. Dans notre malheur, nous avons une chance inouïe : la nature possède une capacité de résilience extraordinaire, proprement incroyable, pour peu qu'on évite d'intervenir. ailleurs, je tiens à attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la France métropolitaine possède la plus grande biodiversité d'Europe. Nulle part ailleurs, ni en Europe ni dans le monde, on ne peut observer, en parcourant un même département, autant de paysages variés. Nous devons faire en sorte que cette richesse 5 000 espèces différentes de plantes, alors qu'il en existe moins de 3 000 en Grande-Bretagne et autour de 2 000 en Pologne. Sur les 114 espèces de libellules dénombrées en Europe, 100 sont présentes en France. Ce sont nos terroirs, qui sont nés de notre histoire géologique, de la fragmentation lors des précédentes glaciations, qui ont créé des foyers d'endémisme à l'origine de cette fabuleuse biodiversité. Aussi profitons-nous d'un foisonnement d'espèces. Je citerai, par exemple, le goujon occitan, le goujon d'Auvergne, le goujon d'Adour malgré cette fabuleuse biodiversité, seulement 1 % de notre territoire national est protégé par des parcs ou des réserves- et encore, il y a de nombreuses dérogations. En Italie, 10 % du territoire national est protégé. Nos voisins européens, même avec des territoires plus petits, plus denses en population, connaissent un plein essor de la faune sauvage, marquant une reconquête bénéfique sans précédent

les phoques gris sont 120 000 en Grande-Bretagne et 500 en France ... Les exemples sont légion. Nous sommes en retard. L'équation est la suivante : nous avons une très grande biodiversité, la plus grande en Europe, spécifiquement française, mais une faune sauvage très en deçà de ce qu'elle pourrait et devrait être, et qui compte également des espèces menacées. La solution est évidente : protéger plus, prélever moins. Il est donc temps, après l'immense avancée de la loi de 1976, d'aller de l'avant, en conscience, en responsabilité.

mes chers collègues, en matière de biodiversité, rien n'égale la Guyane. Ce territoire amazonien compte une immense forêt de 5,3 millions d'hectares et présente une biodiversité exceptionnellement riche, faisant partie des écosystèmes les plus importants au monde avec 5 500 espèces végétales, 684 espèces d'oiseaux, 177 espèces de mammifères et plus de 500 espèces de poissons. Le paradoxe est établi en voyant l'indigence des moyens que l'État, acteur décisionnel, affecte à l'étude de cette biodiversité. Néanmoins, je salue la création de l'agence régionale de la biodiversité de la Guyane, première entité régionale installée en juillet 2018- soit, deux ans après l'Agence française de la biodiversité -et dont on espère la poursuite des missions sans entrave de la part du nouvel office français de la biodiversité. En effet, cette agence contribue d'ores et déjà à la structuration de filières locales en matière de faune et de flore. À cet égard, permettez-moi de mettre en garde contre une transposition à la Guyane de dispositions qui ne lui sont pas adaptées. adaptées. Lorsqu'on parle de faune, notamment sauvage, on parle aussi de chasse. Et sur cette thématique, je rejoins mon collègue Antoine Karam, qui souhaite des dispositions particulières pour la chasse en Guyane, eu égard à l'existence de longues traditions locales ininterrompues et bien établies sur le territoire. En effet, la conception de la chasse en Guyane diverge de celle de l'Hexagone, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'une chasse de loisir, mais, pour bon nombre, d'une chasse vivrière, ancrée dans des pratiques ancestrales raisonnées et nécessaires à la survie de populations occupant le territoire. Les chasseurs de Guyane jouent d'ailleurs un rôle social incontournable dans le cadre du maintien de la biodiversité et de la connaissance de la faune en contribuant à l'aménagement des espaces naturels et des lieux de vie des espèces. ils sont de véritables gestionnaires de la protection de la nature. C'est à ce titre qu'ils mériteraient d'être entendus dans leurs revendications. Ce faisant, la législation cynégétique hexagonale,

Il faudrait que ce projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité maintienne l'équilibre existant et évite un choc des cultures. C'est la raison pour laquelle je soutiendrai les amendements présentés par mon collègue Antoine Karam qui s'inscrivent dans la droite ligne des travaux produits lors des assises de la chasse en Guyane. mon cher collègue. ... il faudrait éviter que, pour des raisons liées à la préservation de la biodiversité, on ne mette la forêt guyanaise sous cloche, créant un « écolonialisme » qui entraverait un développement économique devenu urgent en raison d'une expansion démographique inégalée qui ne pourra plus être ignorée dans un avenir proche. La

Nous précisions ainsi que cette mission incluait le contrôle de la collecte, la centralisation, le traitement de la valorisation des données relatives à tous les prélèvements des espèces chassables. Du coup, on ne comprend pas bien quelle serait la charge financière supplémentaire. Cela devient- hélas ! -une question récurrente. Je prends donc la parole pour insister, à l'occasion de l'examen de cet article 1, sur la nécessité de préciser en toutes lettres dans la loi la mission de contrôle de la collecte et de centralisation, par l'office, des données relatives à l'état de la faune sauvage, et notamment en matière de prélèvements. d'un point essentiel. À défaut, les missions de l'office deviennent caduques. Comment protéger la biodiversité, comment réguler les activités de chasse, si l'on ne connaît pas l'état de la faune dans notre pays ? Dans les faits, contrairement à nos voisins, la France est pour l'instant incapable de produire ces données. Les chasseurs sont censés tenir le compte de leurs prélèvements et transmettre les données à la Fédération nationale des chasseurs, qui agit trop souvent comme une boîte noire dont rien ne sort, ou presque. En conséquence, l'ONCFS produit des estimations hautement imparfaites et sporadiques de l'état de la biodiversité. Ainsi, la dernière enquête date de 2016 et concerne la saison de chasse 2013-2014. La gestion adaptative consiste à chasser de manière durable, en s'autorisant à prélever sans porter atteinte à l'état maximal de conservation de chaque espèce. C'est ainsi qu'elle est pratiquée en Amérique du Nord. Pour connaître les quotas acceptables, il faut suivre les prélèvements sur le long terme afin d'évaluer finement non seulement l'état de conservation, mais surtout l'évolution des populations. Les pêcheurs fournissent des chiffres de prélèvements. C'est ainsi que l'on peut décider de limiter ou de stopper la pêche au thon. Pourquoi ne pourrait-on appliquer ces mêmes pratiques à la chasse ?

Or il manquait déjà plusieurs millions d'euros- environ 200 -à l'AFB pour lui permettre de mener à bien les missions qui lui avaient été confiées par la loi de 2016. La plupart des ressources de ces deux établissements provenaient des agences de l'eau. Il semble utile de rappeler de rappeler que l'État a demandé à ces agences, en 2018, de prendre une part active dans le combat pour la biodiversité en finançant le budget de l'AFB à hauteur de 260 millions d'euros et en donnant 37 millions d'euros à l'ONCFS. Il y a donc fort à parier que l'État continue son hold-up sur la politique de l'eau. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, plusieurs amendements plaidaient en faveur de la suppression de cette ponction de l'État sur les agences. Ces résolutions allaient dans le sens des territoires dont les recettes provenant des redevances de l'eau ont toute leur importance et doivent financer en priorité l'eau. Avec la création de l'OFB, ces établissements vont continuer de subir des coupes budgétaires, ce qui est inacceptable. À l'heure où les réseaux d'eau et d'assainissement de nombreuses communes rurales sont obsolètes, le budget des agences de l'eau doit être impérativement consacré en priorité, sinon de façon exclusive, à la politique de l'eau. Mes chers

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, relative au grand débat national, en application de l'article 50-1 de la Constitution. Cette séance s'organisera en deux temps. Après la déclaration du Gouvernement, la parole sera donnée à un orateur de chaque groupe, puis au Premier ministre pour leur répondre. Puis, après une courte suspension, nous procéderons à un débat interactif de trente questions-réponses.

Même si cela peut surprendre, je voudrais commencer par rappeler que ce grand débat national a été l'occasion, pour bon nombre de nos concitoyens,

les maires de France, qui, avec cet esprit républicain qui les caractérise, ont facilité la tenue du débat. Parfois, ils étaient favorables à l'idée du grand débat ; parfois, ils ne l'étaient pas.

Ils ont évoqué les difficultés qu'ils rencontraient dans l'exercice de leur mission, difficultés que nous devons entendre si nous voulons répondre à celles de nos concitoyens. Je voudrais également adresser aux élus municipaux qui ont dû faire face, samedi après samedi,

transférer la tension des ronds-points dans les salles municipales, ce qui aurait été la pire des choses à faire. J'observe, mesdames, messieurs les sénateurs, en m'en réjouissant, que nos concitoyens ont su,

Avec près de 1,5 million de participants, ce grand débat s'est apparenté à un exercice inédit. Quels que soient nos accords ou nos désaccords, nous pouvons saluer ensemble l'image d'une démocratie vivante, innovante et respectueuse.

Les causes en sont nombreuses. La première, c'est la baisse du pouvoir d'achat de nombre de nos concitoyens depuis la crise financière de 2008,

s'est accrue, le chômage a progressé, la croissance a stagné et les impôts n'ont cessé d'augmenter.

que les inégalités s'accroissent, se figent et se transmettent, que la réussite de leurs enfants dépend plus du milieu de naissance ou du lieu de résidence que des mérites propres de chacun et que, à l'égalité des chances, notre société aurait peu à peu substitué l'inégalité des destins.

pas toute la réalité du phénomène. Il s'agit d'un éloignement géographique, bien sûr, parce que, ici ou là, des lignes de train ont fermé ; ici ou là, des routes estimées nécessaires n'ont pas été construites ou là, des médecins n'ont pas été remplacés ; ici ou là, des services publics ont été fermés ou ont déménagé. Enfin, nos modes de vie, nos règles d'urbanisme,

aux États-Unis. Parce que ces causes n'ont pas disparu et parce que nous avons engagé un certain nombre de réformes, parfois en suscitant des malentendus ou des oppositions, les Français ont exprimé leur colère.

leur indignation. Nous avons commencé à y répondre en annulant la hausse de la taxe carbone et en corrigeant la hausse de la CSG pour les retraités modestes. également pris des mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat, pour que le travail paie davantage. Mais nous avons été au-delà : le Président de la République nous a demandé de prendre le risque d'organiser ce débat, expliquer ce que nous faisions, pour rendre des comptes sur le terrain et offrir aux Français la possibilité inédite de s'exprimer dans ces conditions. Le grand débat a permis de mettre en lumière un certain nombre de vérités. Avant de les évoquer, permettez-moi de m'arrêter quelques secondes sur l'exercice de restitution qui s'est tenu lundi matin. Dans le rapport qu'ils ont publié hier, les garants ont indiqué que cette restitution avait été « fidèle et loyale ». Cette fidélité et cette loyauté nous permettent d'identifier dans ces matériaux d'une très grande richesse les préoccupations et les attentes de nos concitoyens et de les apprécier dans leurs nuances, ce qui nous aidera à placer le curseur au bon endroit pour répondre à des questions

l'incitation ? Jusqu'à quel point devons-nous numériser les services publics ? Comment pouvons-nous revivifier nos outils démocratiques ? Les Français ont joué le jeu du grand débat et, par sa qualité, la restitution donne tout son sens, toute son utilité, à leur engagement. Je le disais, ce grand débat a permis de faire ressortir un certain nombre de vérités. Je pense notamment à l'exaspération fiscale qui a gagné notre pays. Je serai très clair, mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque je parle d'exaspération fiscale ou de ras-le-bol fiscal, pas référence au consentement à l'impôt. Les Français savent qu'ils paient des impôts pour financer des biens communs qui sont indispensables.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il faut bien le reconnaître, au cours des dix dernières années, si l'on additionne tous les prélèvements, les pouvoirs publics ont choisi

2007 à 2017. Nous avions conscience de cet état de fait. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu baisser les cotisations salariales. C'est également la raison pour laquelle nous avons engagé la suppression de la taxe d'habitation. Sans doute l'avons-nous fait trop lentement et pas assez clairement. Nous avons corrigé ce qui devait l'être. Je crois que le grand débat nous invite maintenant à aller plus loin dans la baisse des impôts, mais pas à n'importe quel prix. Les Français ont été très clairs s'agissant de la nécessité de ne pas augmenter les impôts et très clairvoyants sur les conditions s'attachant à cette priorité la baisse des impôts ne doit pas s'effectuer au prix du creusement d'une dette qui est en réalité un impôt pour les générations futures.

du basculement du CICE, qui ne sera applicable qu'une seule année. Nous avons réduit, en 2018, les dépenses publiques en volume de 0,3 %, ce qui signifie que, pour la première fois depuis 1970, les dépenses ont progressé moins vite que l'inflation. Nous avons mis en oeuvre cette politique de baisse de la dépense en faisant des choix de politique publique et en les assumant. Tout va bien ! La deuxième vérité, c'est l'engagement des Français en faveur de l'environnement.

Nous conserverons donc l'ambition et changerons la méthode, en nous appuyant sur les très nombreuses initiatives observées dans les territoires. Nous le savons, la transition écologique est très souvent une transition locale. La troisième vérité concerne la manière dont les Français perçoivent leurs institutions et leurs représentants. J'ai parlé hier, à l'Assemblée nationale, d'un mur de défiance

Elle s'enracine aussi dans des pratiques auxquelles les lois sur le financement de la vie politique,

De ce point de vue, le grand débat nous invite d'abord à construire une démocratie plus délibérative, parce qu'on ne peut plus discuter de l'avenir du pays uniquement tous les cinq ans, parce que le temps médiatique, politique et social s'accélère, parce que nos compatriotes veulent du respect et de la considération.

indépendamment des campagnes municipales, certains projets et événements nécessitent la consultation et le débat avec la population. Cette forme de démocratie existe et se développe

Eh oui ! Nous devons également renforcer notre démocratie représentative, en la rendant plus représentative, plus transparente et plus efficace. Nous avions fait des propositions en ce sens dans le cadre du projet de révision constitutionnelle. Je regrette que nous n'ayons pu envoyer un signal fort aux Français dès l'été dernier. il me semble difficile de ne pas entendre le message pour le moins assourdissant que nous adressent nos concitoyens. Le Président de la République y répondra. La quatrième et dernière vérité concerne nos territoires, et je m'attarderai un peu sur cette question. Le grand débat national a aussi été un grand débat local sur la justice territoriale, l'équilibre à l'intérieur de nos territoires, les relations entre les collectivités et le rôle de l'État. Permettez-moi à cet égard d'évoquer avec vous deux paradoxes qui m'ont particulièrement frappé durant ces trois mois. Premier paradoxe, la défiance envers l'État, son action et son organisation, est immense. Toutefois, les Français ne cessent de se tourner vers lui, pour lui demander de garantir toujours plus de droits et pour les protéger.

Pourtant, nous connaissons aujourd'hui une vraie crise de proximité, à laquelle il faut répondre. Durant ces trois mois, les Français ont exprimé des besoins très précis.

Il s'agit tout d'abord de réconcilier les métropoles avec les territoires qui leur sont proches ou un peu plus lointains. Notre pays a réussi l'exploit- c'est une bonne nouvelle -de rééquilibrer la relation entre Paris et ce que l'on appelait

et les autres parties du territoire doit à l'évidence être rééquilibrée ou repensée. Dans certaines régions et certains lieux, ce rééquilibrage est plus naturel. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les études de flux, les études économiques et les études de solidarité. Ces dernières montrent que, dans un certain nombre d'endroits, la relation entre les métropoles et les territoires qui les entourent est plus harmonieuse que dans d'autres. Il est Il est indispensable, me semble-t-il, si nous voulons répondre à la question de la justice territoriale, que nous sachions imaginer des mécanismes, qui, sans remettre en cause la dynamique des métropoles, soient capables de créer et de développer une telle solidarité.

et répétées. Nos concitoyens accordent une prime à la proximité. Plus leurs élus et les fonctionnaires qui font vivre le service public sont proches, plus ils les respectent et leur font confiance. Avec les associations d'élus, nous prendrons des initiatives concernant le fonctionnement des communes et des intercommunalités, l'articulation entre les régions et les départements et le juste équilibre entre l'État central et l'État local. À cet égard, nous devrons également redéployer des fonctionnaires sur le terrain, en leur donnant le pouvoir et les moyens d'agir localement.

C'est d'ailleurs pour cette raison que nous accélérerons tous les chantiers ayant pour but de garantir à nos territoires les services essentiels que j'évoquais. Je pense au développement du très haut débit pour tous d'ici à 2022. Je me trouvais à Mirande, dans le Gers, le 22 mars dernier, pour faire le point sur la couverture numérique de nos territoires. J'avais eu l'occasion d'évoquer devant vous, au mois de décembre dernier, les tronçons de routes nationales que nous avions décidé de mettre en chantier après parfois plusieurs décennies de pause. Je pourrais également citer le plan Action coeur de ville. Je m'arrêterai quelques minutes sur trois sujets qui se sont invités dans le grand débat. l'avenir de notre système de santé. Si la question n'était pas posée en tant que telle, elle s'est imposée, car les Français considèrent à juste titre qu'elle est essentielle. L'angoisse

Dans quel hôpital accoucher ? Le deuxième sujet est la prise en charge de la dépendance- il s'est lui aussi imposé pendant le débat. C'est la question des Ehpad et celle de la formation des personnels soignants.

Les Français nous ont invités à adopter des approches adaptées à la diversité des territoires, qu'il s'agisse des zones rurales ou des quartiers en difficulté. Ils formulent un plaidoyer qui me réjouit, puisqu'il concerne l'apprentissage, que nos concitoyens perçoivent à juste titre comme la meilleure voie d'entrée dans la vie active. messieurs les sénateurs, nous sommes attachés à la contractualisation, aux solutions sur mesure. Depuis mai 2017, nous avons engagé un grand nombre de contrats territorialisés à l'échelle départementale, avec la Nièvre, avec la Creuse, où je me trouvais le 5 avril, avec les Ardennes, avec le territoire Sambre-Avesnois-Thiérache. Nous avons signé deux contrats d'accessibilité avec les régions Pays de la Loire et Bretagne- le pacte breton engage la région dans la voie de la différenciation. Cette différenciation figurait dans le projet de loi de révision constitutionnelle. J'ai la conviction que, si l'on veut répondre aux attentes formulées par nos concitoyens, nous allons devoir faire en sorte que les réponses de l'État, et de l'action publique en général, soient mieux adaptées aux spécificités des territoires. Cela passe- je le disais -par le principe de différenciation, qui était contenu dans le projet de révision constitutionnelle, mais cela passe aussi par la capacité pour l'État, demain, d'accompagner les projets locaux, exactement dans l'esprit de ce que nous avons fait dans la Creuse-

Un deuxième thème a été très peu présent, et ne s'est pas imposé : celui de la défense, du monde et de ses dangers. Il ne s'est pas imposé ; en revanche, lorsque la question a été posée à nos compatriotes de savoir comment ils envisageaient la réduction des dépenses-

tout ce qui permet de mobiliser plus de policiers et de magistrats, et de mettre plus de moyens à la disposition de nos armées, est nécessaire pour notre pays- c'est l'engagement que nous avons pris, et nous n'y renoncerons pas.

à corriger la méthode, à prendre en compte de nouvelles priorités, à changer d'échelle, peut-être à accélérer parfois- nous devons le reconnaître. Sur d'autres points, elles rejoignent des transformations que nous avons engagées. transformations plus claires, ou, en tout cas, nous concentrer sur les mesures les plus efficaces, pour qu'elles puissent bénéficier directement aux Français. Le Président de la République présentera, le moment venu, ces orientations. Il l'a annoncé : les décisions qu'il rendra publiques seront puissantes et concrètes.

Mais passer du consensus sur le diagnostic, ou même du consensus sur l'objectif, aux compromis démocratiques et aux choix qui font les grandes et les bonnes solutions est un exercice délicat. Avec les élus Avec les élus locaux, quand il s'agit de l'avenir de nos territoires, avec les organisations syndicales et patronales, quand il s'agit de faire vivre la démocratie sociale, avec les associations, dont le grand débat a rappelé le rôle essentiel dans notre vie citoyenne, avec le Parlement, bien entendu, car rien ne peut se faire de grand ni de durable sans le respect des institutions, nous ferons en sorte de bâtir ce compromis démocratique qui est indispensable aux réelles et profondes transformations. Nous serons tous jugés sur notre capacité de construire ensemble ces solutions, dont beaucoup devront être sur mesure, dans la continuité de la République contractuelle voulue par le Président de la République. C'est un très grand défi que nous adressent les Français, avec de très grandes attentes et de très grandes exigences.

j'ai l'impression d'avoir plus appris au cours de ces six derniers mois qu'en trente ans de vie publique. Pour tout dire, j'ai aussi entendu plus d'âneries en six mois qu'en trente ans. Et pourtant, Et pourtant, depuis trente ans, nous en avons tous pas mal entendu ! Si, comme disait Talleyrand, la politique est l'art d'agiter les peuples avant de s'en servir, alors nous avons pris une grande leçon de politique de la part de quelques gouverneurs de rond-point, qui ont réussi à transformer en fureur la colère de quelques dizaines de milliers de personnes et à leur faire croire qu'ils sont, à eux seuls, le peuple français. Il ne reste

sur fond de poubelles en feu en répétant « on nelâche rien », sans que l'on sache d'ailleurs ce qu'ilstenaient. Le spectacle est navrant ; et pourtant, beaucoup d'inquiétudes sont réelles. L'objectif du grand débat, si j'ai bien compris, est d'y répondre. Sa principale vertu, c'est qu'il a remplacé les révoltés des braseros, plus centrés sur eux-mêmes qu'un trou noir et refusant tout dialogue, par des élus locaux et leurs concitoyens dans les mairies.

mais l'ébauche seulement, car il reste la profusion et la dispersion des milliers de contributions écrites ou orales. Il reste le fait que beaucoup de propositions entraîneraient, si elles étaient adoptées, un résultat terriblement français : l'explosion des dépenses publiques. La conclusion du grand débat, c'est un peu une lettre au père Noël, et si le président ne veut pas passer pour le père Fouettard, il va devoir réussir à expliquer que la différence entre le grand débat et le Gouvernement, c'est que le Gouvernement ne peut s'affranchir du réel. Et le réel, c'est que nous sommes les champions du monde de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. Emmanuel Macron l'avait expliqué lors de la campagne de 2017, tout comme d'ailleurs son adversaire de la droite républicaine. Ni le constat ni les remèdes n'ont changé depuis. Ils s'appellentréforme des retraites- la vraie de la fonctionpublique, de l'assurance chômage, du code dutravail, de l'éducation et de la formation, urgenceclimatique, etc. Si l'issue du grand débat devaitêtre de l'oublier, de céder à tous ceux qui demandent « des annonces fortes », c'est-à-dire, en clair, encore plus de dépenses, alors tout estperdu. En un mot, le président a promis d'entendrele grand débat- c'est heureux -, mais il va falloir aussi,pour une part, qu'il lui résiste, et qu'il résiste, avant tout, à la désespérante tendance de ce pays à toutattendre de l'État, ce qui ne conduit ni à l'optimismeni à l'initiative. pour preuve les enquêtes qui nousapprennent qu'une majorité des jeunes Français ontpeur de l'avenir, ce qui n'est jamais arrivé nulle partdans l'histoire, pourtant infiniment plus ingrateenvers toutes les générations qui nous ont précédésqu'envers la nôtre. Ce ne sont pas les temps qui sontdevenus plus durs ; c'est nous qui nous sommesamollis. Il y a un autre sujet sur lequel il va nous falloir résister tous ensemble : celui des nuages qui s'amoncellent sur notre démocratie. Les populistes ont tous un point commun : ils prétendent toujours démocratiser la démocratie, rendre le pouvoir au peuple et chasser les élites responsables du mal. Le problème n'est pas français ; il est global. La crise des « gilets jaunes » est la version hexagonale d'un péril qui s'appelle ailleurs Brexit, Salvini, Erdogan ou Bolsonaro. Cette crise est triple : crise de la représentation, crise de la montée de l'impuissance publique et crise du déficit de sens. Elle frappe toutes les démocraties et réjouit les dictatures, qui savourent déjà leur revanche. Elle est aggravée par une technologie numérique dont nous pensions qu'elle serait un formidable outil de dialogue, de transparence, d'information et de raison et qui s'est révélée un redoutable instrument d'intolérance, un cauchemar orwellien dans les pays totalitaires et un déni de la vie privée chez nous, le plus grand vecteur de désinformation jamais inventé et le porteur du pire de l'émotion et de l'indignation. « Nul ne ment autant qu'un homme indigné », disait Nietzsche. Et nous sommes aujourd'hui atteints d'indignationnisme. Et c'est le moment où certains, monsieur le Premier ministre, vous demandent de remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe. Parce qu'on peut aujourd'hui se procurer d'un clic un costume, une voiture d'occasion ou même un partenaire d'un soir, certains pensent que l'on peut faire la loi ou révoquer le président en un clic. Ils ne voient pas que cette démocratie directe, c'est ce que nous avons sous les yeux depuis six mois : la démocratie des réseaux antisociaux, avec, au nombre de, Fly Rider comme président. « La foule est La foule est traître au peuple », disait Victor Hugo, et la démocratie directe proposée par les populistes est le triomphe de la foule. Nous voyons bien, déjà, que derrière le masque avenant du référendum d'initiative citoyenne se cache le visage plein de ressentiment du référendum révocatoire. Je comprends que l'on souhaite une démocratie plus participative, dans cette V République si comment dire ? -jupitérienne. Et il va nous falloir trouver un équilibre. Mais ce n'est pas au moment où tout semble glisser, déraper, devenir incontrôlable, qu'il faut affaiblir la démocratie représentative. Entre Montesquieu et Tocqueville, d'un côté, Drouet et le boxeur du pont des Arts, de l'autre, je choisis les premiers, même s'ils n'ont pas d'amis sur Facebook. Cela m'amène à la réforme constitutionnelle. Le dégagisme a contribué à l'élection du Président de la République. Il en a joué, comme les autres candidats d'ailleurs, en promettant de dégraisser le Parlement- promesse étonnante, quand on sait que la France compte deux fois moins de parlementaires par habitant que la moyenne européenne. Très juste ! Personne n'a dit cette vérité aux Français pendant le grand débat ; dans le cas contraire, l'approbation serait peut-être moins massive. Mais c'est une promesse de campagne, et il est logique de s'attendre à ce que le Gouvernement veuille la tenir. Le président du Sénat l'a bien compris, qui avait accepté le verdict des urnes avec discipline républicaine et avec fermeté, en disant au chef de l'État que le Parlement était prêt à envisager un plan social, mais pas une hécatombe. Les deux n'étaient pas loin de toper. Récemment, j'ai cru comprendre que les relations du Sénat et de l'exécutif s'étaient ... rafraîchies. Je crois que nous sommes tous assez expérimentés pour faire notre examen de conscience réciproque, afin d'éviter une guerre qui, en ces temps de des élus, ne ferait que des victimes. En ce qui me concerne, j'avoue n'avoir pas été transporté par le signalement de hauts fonctionnaires à un procureur. Mais, d'un autre côté, mesdames, messieurs les ministres, ce n'est tout de même pas la faute du Sénat si M. Benalla est le seul éléphant au monde qui se promène avec son propre magasin de porcelaine.

Il faut sortir de cette crise qui fait tant de mal à la France et à son image. Ce sera difficile, parce que nous avons tous compris que le dégagisme ne s'adresse pas qu'aux parlementaires, mais à toute la classe politique, Président de la République compris, à toute l'administration, haute ou pas, et même, pour la première fois, jusqu'à certains élus locaux. Il faut en sortir ensemble, sans démagogie et sans faiblesse ; sinon, c'est ensemble que nous serons balayés par les démagogues et les faibles, par tous ceux qui combattront les réformes courageuses dont la France a besoin et qui soutiendront celles qui continueraient à nous faire plonger. C'est le défi qui nous attend. La

sans enthousiasme, parce que nous savions bien qu'une sortie de crise ne pouvait pas s'opérer uniquement par la voie traditionnelle, rituelle, des concessions financières massives payées par toujours plus d'endettement.

traduisait beaucoup plus qu'une demande de simple amélioration de l'ordinaire. Ce qui était en cause, c'était les perspectives d'existence de chacun

la Nation était profondément divisée. Et elle l'est toujours- tel sera le prochain et principal défi des mois à venir. La seconde proposition consistait dans Je voudrais simplement observer, monsieur le Premier ministre, que l'exercice d'aujourd'hui est un peu vain : nous ne votons sur rien et vous ne nous avez pas proposé de solutions, puisque vous attendez celles de Jupiter.

500 000 contributions, mais certaines copiées-collées. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. Ce sont des contributions de Français, et non pas la contribution des Français : les contributeurs

médiatique, a tourné au monologue. Le Président de la République a très vite confisqué ou monopolisé la parole, au point qu'il semblait dire que le débat c'était lui, lui seul, tombant ainsi dans une ornière qui l'avait déjà précipité dans les difficultés face à ce mouvement spontané des Français. De ce constat, je pense que l'on peut déjà tirer une conclusion en matière démocratique. La démocratie participative est évidemment intéressante, mes chers collègues.

car il y a des paroles qui portent plus que d'autres : certains, certaines minorités, manient mieux la parole que d'autres. Seul le suffrage réalise l'égalité : un homme, une femme, une voix. Exactement Le général de Gaulle avait pour habitude de dire que la parole du peuple est la parole du peuple souverain, celle qui a été, en France, trop souvent contournée, du référendum constitutionnel que d'une consultation publique -de Notre-Dame-des-Landes. Monsieur le Premier ministre, ma conviction est que vous ne soignerez pas la blessure faite à la souveraineté populaire

de peser sur sa destinée et de la maîtriser. C'est la grande question démocratique ! Et je pense, avec beaucoup d'autres, que vous ne pourrez sortir de ce grand malaise sans une consultation nationale.

Il faut refermer très vite ce grand débat : le grand débat a assez duré, et le temps des décisions est enfin arrivé. Mais il n'y aura pas de sortie de crise

que notre économie et nos entreprises ne créent pas suffisamment de richesses, parce qu'elles ne sont pas suffisamment compétitives, pour améliorer durablement leur niveau de vie. Nous devrons leur dire qu'il faudra mettre plus de travail sur la table si nous voulons préserver un modèle social

Mais il ne suffira pas de dire que les Français paient trop d'impôts. Il va falloir dire maintenant quelles sont les dépenses publiques qu'il faut baisser, parce qu'il n'y aura pas

Jamais les collectivités n'ont, pour les compétences qui leur ont été attribuées, disposé de si peu de moyens ! Jamais en France il n'y a eu de révision si autoritaire des structures territoriales : le grand remembrement

Il va falloir en tirer les conséquences, des conséquences radicales sur la décentralisation, sur les compétences, sur les niveaux de subsidiarité, mais aussi sur l'action de l'État.

Parlera-t-il longtemps ? Peut-être ... Nous lui reconnaissons une forme de résistance. Mais parlera-t-il clair ? Parlera-t-il vrai ? Sans courage de dire, il n'y a pas de courage de faire. Je pense que les Français en ont marre des subtilités, des habiletés, des ruses, du « en même temps », d'une « pensée complexe ». Ce qu'ils veulent, c'est non pas de la complexité, mais de la clarté à l'égard d'une vision de l'avenir,

au nom de la République et au nom de la France

Jamais les Français ne se sont autant pris à discuter, à argumenter, à échanger, à débattre, à se rassembler autour du bien commun. Oui, mes chers collègues, les citoyens français font honneur à notre pays lorsqu'ils se saisissent de leur avenir En apportant leur pierre à l'édifice de notre idéal républicain, ils ont prouvé à tous leur volonté de ne pas baisser les bras. Ce n'est pas une surprise : les Français sont coutumiers du fait. Ils ne se dérobent pas devant l'Histoire. Ils n'évitent pas le débat. Partout, ils se rencontrent. Partout, ils s'en emparent. Le grand débat, n'en déplaise à certains, a été utile et fécond. Douze milliards d'euros ... Il a donné les moyens aux Français de s'exprimer sur la situation du pays, sur les grands enjeux de notre avenir, comme sur les difficultés du quotidien. est un succès de participation ; vous l'avez rappelé. C'est aussi un succès de propositions. Les Français se sont exprimés en toute liberté. Ils se sont largement mobilisés. Nombreux

Chacun a son analyse de la crise que nous vivons. Certains pensent que le malaise exprimé, la défiance à l'égard de toute forme de pouvoir et le procès en illégitimité des dirigeants sont dus à la politique de l'actuel gouvernement. gouvernement. Ceux-là font preuve d'une amnésie, d'une hypocrisie et d'une cécité qui laissent bien peu de place à la modestie et au devoir de responsabilité, alors que cette crise- chacun le reconnaît

les principales attentes évoquées à l'occasion de ce grand débat ? Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit hier, les Français attendent de la justice, une plus grande défense de l'intérêt général et de l'efficacité ; j'y souscris totalement. Ils souhaitent une juste affectation de l'argent public, une juste contrepartie de leurs efforts envers la collectivité. Ils comprennent que chacun doit oeuvrer dans le sens de l'intérêt général, à commencer par ceux qui ont un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire nous-mêmes. L'intérêt général n'est pas la somme d'intérêts particuliers ; il doit guider l'action de chacun. C'est l'efficacité de l'action publique qui est en jeu. Je pense notamment à la lutte contre les inégalités scolaires, au taux de chômage, encore trop élevé, ou à la désertification médicale, pour prendre quelques exemples. Ce sont les promesses non tenues qui alimentent une rancoeur exprimée en grogne permanente, explosant parfois en bouffées de colère. C'est une revendication quotidienne. Nous devons y répondre. C'est pourquoi le Gouvernement tient ses engagements. Si nous devons faire davantage, beaucoup a déjà été fait ; je l'ai souligné. S'il y a une impatience quant aux résultats, chacun ici sait bien que les meilleures réformes et les meilleures lois n'agissent pas dans l'instant, comme le feraient croire les incantations de magiciens sans scrupules. Pour retrouver la confiance, il faut apporter des réponses aux trois exigences qui émergent des consultations : la justice fiscale, la justice sociale et la justice territoriale. La demande de justice fiscale est un sentiment normal face à un système complexe et parfois illisible. C'est pourquoi le Gouvernement et sa majorité se sont engagés sur des mesures fortes : la suppression de la taxe d'habitation, qui représente plus de 20 milliards d'euros. La justice fiscale, c'est aussi la taxe GAFA, sur les géants du numérique. C'est également la suppression des cotisations sociales salariales d'un montant de 4 milliards d'euros. Pourtant, la classe moyenne nous dit C'est nous qui payons pour tout le monde. » Elle s'interroge : « Où va donc l'impôt ? » C'est en l'orientant vers elle que l'action de l'État prendra tout son sens. La France est le pays qui redistribue le plus, et les Français ne le ressentent pas. D'où vient cette incompréhension ? Il faudra aussi y apporter des réponses. Le Gouvernement entend baisser les impôts. Il le fait déjà. Pour qui ? Pour les entreprises, pour créer de l'emploi ; pour les ménages, pour le pouvoir d'achat. Cessons de penser que l'on peut toujours dépenser plus sans jamais économiser ; oui, monsieur Retailleau, vous avez raison de le dire Les Français ont aussi exprimé une demande forte de justice sociale. D'où la suppression de l'ISF ? Le Gouvernement a lancé le plan pauvreté, pour un milliard d'euros. Cette exigence se retrouve aussi à travers l'investissement dans l'apprentissage, la formation et l'insertion. Et ne l'oublions pas, lutter contre la pauvreté, c'est d'abord lutter contre le chômage. C'est l'action première que mène le Gouvernement depuis deux ans. Enfin, les Français réclament avec force l'urgence d'une justice territoriale. Nous sommes, au Sénat, les premiers observateurs de la montée de nouvelles inégalités et d'une fracture entre la France rurale et la France urbaine, source de marginalisation et d'isolement. Là, nous devons aller plus loin, monsieur le Premier ministre. Une première étape a été franchie avec des dotations de fonctionnement stabilisées, des dotations d'investissement augmentées et des clés données aux administrations pour adapter leur action aux territoires. Mais pas aux élus ! Il faut redéfinir le lien entre les communes et l'intercommunalité et rouvrir intelligemment le chantier de la loi du nous avons entendu l'engagement et la fermeté du Gouvernement pour répondre à ces urgences. Nous devons poursuivre les réformes pour que l'action aboutisse. Oui à la baisse des impôts

comment interpréter- vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre -des injonctions contradictoires ? Plus de proximité, et moins d'élus ; des économies sur la défense et le logement, alors que l'urgence sécuritaire et le besoin de logements n'ont jamais été aussi flagrants et primordiaux. Si les Français ressentent que les injustices se creusent, il faut mieux indiquer le sens des mesures qui sont prises pour y remédier. Monsieur le Premier ministre, nous avons perçu votre capacité d'écoute et votre détermination à répondre aux attentes des Français.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, marquée, au-delà du « tout pour la finance », par le choix d'un libéralisme sans frein, de la casse du droit du travail à la sélection renforcée pour entrer à l'université en passant par la déstructuration de la SNCF, semblait, coup après coup, consolider un grand fatalisme, une sensation que, dans un paysage politique explosé, la résistance ne pouvait pas s'organiser. La voie semblait libre pour les apprentis sorciers du CAC40, ces partisans d'un nouveau monde sans droits, sauf pour les plus forts. Mais l'attitude jupitérienne du Président de la République, son arrogance et son jusqu'au-boutisme libéral, symbolisé par la suppression de l'ISF, ont provoqué l'explosion de la colère populaire qui s'exprime depuis maintenant cinq mois. Les discours sans fin, les « en même temps » permanents et les petites phrases méprisantes à l'égard du peuple ont accompagné cette politique de démolition méthodique des derniers vestiges du modèle social français issu du programme du Conseil national de la Résistance. Depuis des décennies, la solidarité recule en France. Les droits les plus fondamentaux, pourtant reconnus par la Constitution, comme le droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé, à l'éducation ou à une retraite digne, sont sont aujourd'hui bafoués. Des décennies de renoncement ont amené à la profonde crise économique et sociale, mais aussi démocratique, que connaît notre pays, comme l'ensemble du monde occidental. La clé du renoncement, l'alpha et l'oméga du libéralisme, c'est la primauté de l'argent sur l'être humain. Élu Président de la République, Emmanuel Macron a prôné un « nouveau monde », qui, bien vite, est apparu pour ce qu'il est un régime libéral à l'autoritarisme croissant, usant et abusant de « coups de com' » pour masquer les grands bonds en arrière sur le plan social et économique. La colère est venue. Elle a éclaté. Depuis vingt et une semaines, la France vit au rythme du mouvement social et citoyen le plus long de son histoire. La longueur de cette secousse souligne la profondeur de la souffrance. Vous avez peiné, monsieur le Premier ministre, à juguler la violence qui, inévitablement, accompagne ces colères. Aux actes illégaux de quelques-uns, que nous avons condamnés avec force, vous avez répondu par une répression systématique et démesurée du mouvement. Jamais Jamais vous n'évoquez ces centaines de blessés, ces dizaines de mutilés et d'éborgnés. « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » écrivait le poète. Est-ce ainsi que ceux qui relèvent la tête, ceux qui osent dire « non » doivent être considérés ? être considérés ? Cette violence, vous ne l'avez pas évoquée, même d'un souffle, ni au Grand Palais ni ici, à mille lieues des ronds-points. Ce grand débat, monsieur le Premier ministre, n'est pas celui de nos concitoyens. Tous les chiffres le montrent. Sur 45 millions d'électeurs inscrits, auxquels s'ajoutent des millions de jeunes en mesure de comprendre et d'agir, comme ils le font sur le climat, seuls 500 000 personnes, soit 1 % à peine du corps électoral, ont élaboré des contributions, ce chiffre étant lui-même fortement contesté. Et 1,5 million de personnes auraient participé à des débats, ce chiffre n'étant pas contrôlable. Quant aux conférences régionales, à neuf Français sur dix tirés au sort ont refusé d'y participer. Pourtant, ce grand débat aurait pu rassembler et être autre chose qu'une tentative de contournement de la colère populaire. Mais Emmanuel Macron a dès le départ écarté les thèmes de justice sociale et de justice fiscale qui fondaient la mobilisation : pas question de rétablir l'ISF ; pas question d'augmenter le SMIC

de l'expression populaire. Je ne suis pas née de la dernière pluie, mais quand même ... L'opération à laquelle nous assistons- faire passer ce grand débat pour l'expression du peuple -est sidérante. « Plus c'est gros, plus ça passe » pourrait être votre adage et celui de M. Macron. Bravo ! La France qui souffre,

La belle photographie que vous voulez nous vendre comme une reproduction parfaite pour légitimer votre fuite en avant libérale est totalement faussée. La preuve : alors que 77 % des Français demandent le rétablissement de l'ISF, 10,3 % des contributeurs au grand débat y seraient favorables 90 % des sondés souhaitent un abaissement de la TVA sur les produits de première nécessité contre 13 % seulement des contributeurs ; plus de 80 % des Français sont favorables au RIC contre 5,8 % des contributeurs. Quel décalage ! Ces chiffres montrent bien que ce grand débat tourne à la grande entourloupe. Très bien ! Emmanuel Macron et vous-même prenez un grand risque. Non seulement vous tentez une grossière manipulation pour justifier le non-reniement et un entêtement dangereux, mais vous masquez la poursuite des coups bas contre les intérêts populaires, semaine après semaine, mois après mois. Quelle hypocrisie à parler d'écoute alors que vous vous obstinez à brader au privé Aéroport de Paris, ADP, et la Française des jeux Écoutez le peuple, et une bonne fois pour toutes ! Si vous avez un doute sur ADP, acceptez le référendum ! Pourquoi quelques conseillers financiers ou grands argentiers auraient-ils raison face à la volonté de millions de femmes et d'hommes ? Avec les 240 premiers parlementaires signataires de la proposition de loi référendaire, je mets au défi Emmanuel Macron de lancer une telle consultation populaire. De même, vous affirmez avec des trémolos dans la voix la nécessité de rapprocher les services publics de la population. Mais, monsieur le Premier ministre, vous venez de déposer un projet de démolition du statut de la fonction publique en confirmant la suppression de 120 000 fonctionnaires. Et vous asphyxiez toujours et encore les collectivités locales. C'est la même logique avec votre annonce d'une augmentation de 5,6 % de l'électricité dès cet été. Monsieur le Premier ministre, le piège s'est refermé sur vous. Si, si ! Pour appliquer le programme d'Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas répondre aux attentes populaires, populaires, tout simplement parce que votre logiciel politique est incompatible avec les espoirs de nos concitoyens. J'en veux pour preuve que la petite musique de la nécessaire réduction des dépenses publiques est déjà là. là. Mais jamais vous n'évoquez la scandaleuse évasion fiscale et l'enrichissement sans fin des détenteurs de capitaux. C'est logique : vous êtes là pour les servir ; ce sont vos soutiens indéfectibles. Vous maquillez le désir de justice fiscale en volonté de baisse des impôts et avant tout pour les plus riches et les entreprises. Quant à la justice sociale, salaires ou retraites, seule votre règle d'or, celle de l'austérité, prévaut. Monsieur le Premier ministre, avec Emmanuel Macron, vous prenez le risque de multiplier la colère. Ces derniers mois montrent que l'histoire n'est pas écrite. Vous prenez le risque non seulement de décevoir, mais aussi de susciter le désarroi pire, de susciter la haine ! L'Histoire aurait pu retenir le souvenir d'un pouvoir qui aurait choisi l'écoute et la raison. Malheureusement, tout montre que vous vous apprêtez à faire le choix de l'entêtement, celui des privilèges au détriment de l'humain, de cette humanité qui a forgé dans les épreuves l'histoire de notre pays. Il faut conclure, ma chère collègue.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre pays a connu ces derniers mois deux phénomènes inédits : d'abord, les « gilets jaunes » ; puis, le grand débat. Ces deux moments sont liés entre eux et indissociables sans les « gilets jaunes », qu'il ne faut pas mépriser, il n'y aurait pas eu de dialogue avec les Français. Je veux d'abord saluer ce moment qu'a été le grand débat. Un risque a été pris de qualifier de « grand » un débat qui n'avait pas encore eu lieu. Mais il faut reconnaître aux Français leur goût de la démocratie, leur plaisir à débattre, leur volonté de se faire entendre. Nous regrettons suffisamment l'abstention aux élections pour ne pas saluer cette envie de proposer dans le cadre du grand débat. socialistes, partageons ce sens démocratique du débat. C'est pour cette raison que nous avons participé dans nos territoires aux réunions qui s'organisaient. C'est dans cette même philosophie que nous avons répondu aux invitations officielles du Président de la République lors de sa tournée médiatique en seize dates. C'est aussi dans cet état d'esprit que nos sénatrices et sénateurs représentant les Français établis hors de France ont organisé partout dans le monde une consultation auprès de nos concitoyens, recueillant plus de 16 500 réponses remises au Gouvernement, et dont les premiers éléments font ressortir des préoccupations similaires à celles Seulement, monsieur le Premier ministre, ce débat aurait pu ne jamais avoir lieu. Si vous l'avez organisé, c'est sous la contrainte ; il faut bien le rappeler. Sans les « gilets jaunes », il n'y aurait pas eu davantage les mesures annoncées le 10 décembre. Sans cette poussée de fièvre des Français, la taxe carbone serait toujours en place. Eh oui ! Les retraités qui touchent moins de 2 000 euros paieraient encore la CSG au prix fort. Exactement ! Des centaines de milliers de Français n'auraient pas bénéficié du coup de pouce à la prime d'activité. Tous ces changements dans votre politique étaient pourtant réclamés depuis des mois sur les travées de gauche et par de nombreux syndicats. Ces mesures, bien qu'insuffisantes, notamment parce que vous n'êtes pas revenu

Il aura fallu que les Français vous les arrachent. Nous sommes donc à un moment charnière aujourd'hui. Les 10 milliards d'euros du mois de décembre, d'ailleurs essentiellement financés par la solidarité nationale et très peu par les employeurs, ont permis de traiter quelques symptômes sans guérir le pays de toutes les injustices de votre politique. Le grand débat a fait office de palliatif au manque d'écoute de ce début de quinquennat- vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même -sans mettre un terme à la fièvre et à la colère d'une France abandonnée. Cette France attend désormais des réponses. Allez-vous la décevoir ? Car le constat du grand débat est posé. Notre pays subit une fracture sociale à cause de la crise du pouvoir d'achat et de la diminution des services publics. Ce que vous refusez d'entendre, c'est la demande des Français d'avoir accès à des services publics performants, partout performants, partout sur le territoire. Ce besoin est renforcé par les fractures dans l'emploi, liées au chômage notamment. Le tout aggravé par des fractures territoriales du fait des différences géographiques, qui se creusent, et du sentiment d'éloignement, qui s'accroît. Ces évolutions de la société en viennent à isoler encore plus les familles monoparentales, les personnes seules ou âgées et les Français qui sont éloignés des grands centres urbains. Face à ce constat, la question peut être résumée ainsi : comment redonner confiance aux Français alors que votre politique a perdu toute crédibilité ? Nous vous avions fait une proposition pour y répondre : organiser une grande conférence sociale, environnementale et territoriale pour traiter et trier ce qui est remonté du terrain avant de décider.

sont celles d'Emmanuel Macron, qui est en même temps le sélectionneur, l'arbitre, le gardien de but, l'avant-centre et le commentateur. C'est une raison supplémentaire qui devrait vous pousser dans les bras des corps intermédiaires pour mieux agir, ce que nous ne voyons toujours pas. Écoutez-nous, monsieur le Premier ministre ; personne dans cet hémicycle n'a intérêt à ce que vos conclusions provoquent une nouvelle crise sociale, en confondant ce que vous souhaitez décider et ce qui est réellement remonté des Français. Écoutez-nous, car, comme sur la privatisation d'ADP, vous ne pouvez pas toujours avoir raison tout seul, tout le temps et contre tout le monde Malheureusement, nous avons peur, à vous entendre, que vos choix ne soient déjà faits depuis des semaines. Si le Président de la République a peut-être gagné un peu de temps, j'espère qu'il ne nous a pas fait perdre le nôtre. les sujets qui sont remontés figure tout d'abord la question des services publics. Dès le départ, nous avons estimé que votre questionnaire était extrêmement mal posé, voire orienté, le service public n'étant interrogé que sous le prisme du coût budgétaire et des économies à réaliser, jamais sous celui de l'intérêt social, économique et environnemental. Le débat a permis de révéler aux yeux de tous combien le désert des services publics dans notre pays était central dans les préoccupations de nos compatriotes, provoquant même souvent ce sentiment d'abandon que chacun a pu commenter. Cela fait des années que cette problématique est évoquée, mais nous devons bien remarquer cette tendance de fond à la disparition des services publics dans les zones éloignées des grands centres. Il est urgent de rompre avec une telle logique, d'abord guidée par des préoccupations budgétaires court-termistes. Pour nous, le service public est au contraire ce qui permettra de retisser les liens d'une société fracturée et malmenée. La question des services de santé, particulièrement des maternités, a animé les réunions dans de nombreux départements. Je veux notamment évoquer ici les outre-mer, territoires trop souvent oubliés, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur l'accès aux soins. Il est urgent d'inverser le processus de disparition des établissements de santé et de réimplanter dans tous les territoires un accès aux urgences, aux maternités et aux soins quotidiens. Lorsque nous constatons sur un plan statistique que l'éloignement et le faible accès médical augmentent les risques de santé, il est déjà trop tard. J'ai pris l'exemple de la santé, mais j'aurais pu évoquer aussi les mobilités, l'accès à une justice pour tous les Français ou l'éducation, qui sont synonymes de puissance publique, de puissance publique, pas de désengagement budgétaire. C'est sans doute là que nos points de vue divergent. Oui, les services publics ont un coût ! Mais nous disons également qu'ils ont une valeur De la même manière, vous ne pouvez pas expliquer aux Français que vous voulez réaliser des économies en raison de l'accès aux services publics au travers de plateformes électroniques. Savez-vous combien de Français n'ont toujours pas accès à internet ou ne bénéficient pas d'une couverture digne de ce nom ? En raisonnant comme cela, vous aggravez la fracture entre nos concitoyens Le besoin de plus de proximité est, selon nous, un des enseignements premiers du débat, sur tous les plans, y compris le plan démocratique. Nous voulons nous faire ici les porte-voix de ceux qui, parmi nos concitoyens et les élus locaux, ont exprimé le besoin d'une meilleure répartition des pouvoirs dans notre pays. Cette vision de redistribution des pouvoirs a deux faces. La première est celle de la décentralisation, avec un nouvel acte attendu qui redonnerait des compétences et des moyens d'action, notamment budgétaires, aux élus locaux. Donnons aux collectivités un pouvoir accru de fiscalité. Décentralisons notre économie les régions. Donnons des capacités d'investissements dans le logement et les infrastructures de mobilité, y compris aux communes, aux communes, sans oublier les très grands projets structurants : permettez-moi d'évoquer le canal Seine-Nord Europe, pour lequel nous n'avons toujours pas de certitude quant au financement de l'État. Défendons aussi la capacité de formation et de soutien à l'apprentissage dans les collectivités et par les collectivités ; vous avez vous-même prôné cette l'Assemblée nationale, en contradiction avec la loi que vous avez fait voter l'été dernier. Notre objectif de décentralisation s'oppose à votre souhait de contractualisation, qui est le projet d'un État toujours plus centralisé qui ne fait pas confiance à l'intelligence des élus locaux. La deuxième face de la décentralisation, c'est la redistribution des pouvoirs entre les citoyens. Même si nous pensons que la démocratie représentative est le système le plus équilibré pour faire face aux crises, notre démocratie est aussi mûre pour mieux impliquer nos concitoyens dans les décisions, qu'elles soient nationales ou locales. Les mécanismes de consultation et d'interpellation existent et ne passent pas forcément par le référendum à caractère binaire. Nous avons déjà fait des propositions en ce sens dans le cadre du débat constitutionnel. Cette démocratie décentralisée est pour nous exclusive des fausses solutions que sont la réduction du nombre de parlementaires, la recréation du conseiller territorial sans réflexion sur l'organisation préalable des collectivités, l'affaiblissement du bicamérisme. Ces propositions aventureuses n'apporteraient rien de mieux à notre démocratie, bien au contraire, puisqu'elles réduiraient encore un peu plus la place des élus et des citoyens face aux administrations centrales ! Enfin, j'en viens à mon troisième thème, qui préoccupe notre siècle, celui de l'écologie. Notre époque doit prendre des décisions fondamentales pour les prochaines générations. Ce poids de la décision ne doit plus nous tétaniser. C'est le sens du message envoyé par les grands absents du débat, que sont les jeunes de notre pays. Plutôt que de venir s'exprimer dans un débat trop peu centré sur ces questions, ils ont préféré battre le pavé à leur tour ! Nous devons entendre, nous devons agir pour transformer notre économie, pour plus de coopération et moins d'émissions carboniques. Là encore, l'Europe est à mobiliser, en soustrayant les investissements écologiques des critères de déficit pour que notre pays puisse, enfin, adapter sa production et sa consommation d'énergie. En matière de protection de l'environnement, les technologies existent, les moyens existent, le soutien populaire existe. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique, votre volonté politique, monsieur le Premier ministre ! C'est, bien sûr, sur ce sujet que vous serez le plus attendu, particulièrement par la jeunesse de notre pays. J'aurais pu aborder bien d'autres sujets qui ont structuré ce grand débat, celui du logement qui pèse de plus en plus dans le portefeuille des ménages par manque de soutien public, celui de la justice fiscale que vous confondez avec la baisse générale de la fiscalité. Vous continuerez à nous trouver pour demander le rétablissement de l'ISF et à nous trouver aussi pour que cette contribution soit mise à jour au profit de nos concitoyens. Très bien ! Monsieur le Premier ministre, un jour, nous ferons le bilan des mauvaises mesures fiscales qui ont été les vôtres au début du quinquennat. j'aurais pu aborder le sujet des salaires dont la stagnation durable mériterait une conférence salariale urgente entre syndicats et patronat. Ces trois axes, logement, justice fiscale et niveau des salaires, sont pour nous les trois composantes de la question centrale de ce débat. trois leviers qu'il faut appuyer, sans se limiter à la baisse indifférenciée des impôts, qui exprime une vision simpliste, de court terme. Elle profitera toujours à ceux qui ont les moyens et n'enrayera pas la pauvreté

C'est pour cette raison que vous devez aujourd'hui apaiser, monsieur le Premier ministre, en vous appuyant sur tous les partenaires sociaux, collectivités, élus, pour que le débat ne reste pas sans lendemain et pour que la confiance soit retrouvée. Je voudrais vous le dire très simplement, monsieur le Premier ministre, votre politique, vos dits et vos non-dits restent anxiogènes, anxiogènes pour l'âge de la retraite et sa fixation, anxiogènes pour le statut des cinq millions et demi de fonctionnaires, anxiogènes pour les ressources des collectivités locales, anxiogènes pour nos libertés publiques, anxiogènes pour la préservation de la loi de 1905, anxiogènes pour le financement des aides au logement. En un mot, je voudrais ainsi utiliser vos propres termes pour résumer un message de ce débat continuez d'écouter, pour bien entendre, et sachez entendre ! Pour qu'il y ait de la paix sociale dans ce pays, il faut aussi de la justice sociale

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, le temps de la démocratie n'est certainement pas celui des médias.

Bien au contraire, notre République se nourrit du principe fondamental selon lequel la volonté générale s'exprime à la fois par la voix du peuple souverain et par celle de ses représentants. Cette construction politique, héritage de notre histoire, garde toute sa force à l'heure où les populismes veulent nous imposer leur idéologie mortifère. Or nous avons vécu ces derniers mois au rythme des samedis de manifestations, puis de violences intolérables. Nous avons subi l'irresponsabilité de certains médias, pour qui le sensationnel fait figure de ligne éditoriale, au risque d'attiser des feux qui ne demandaient qu'à s'embraser. Nous avons subi la lie de la désinformation, des rumeurs, pointant du doigt une catégorie de population, défiant la raison que nous tenons des Lumières, provoquant même parfois des réactions collectives que nous pensions réservées aux périodes obscurantistes. Il est certain que ce que traverse notre pays doit inciter à la retenue et à la modestie. De façon plus générale, il souffle en Occident des vents mauvais qui veulent détruire l'héritage des Lumières. Ce qui se passe aux États-Unis, en Italie, en Pologne, en Hongrie nous concerne directement. Le devenir de l'Union européenne en est à un moment clé, qui exige que nous soyons collectivement responsables. Oui, des colères se sont exprimées, parfois avec véhémence. C'est le propre d'une démocratie ! Parfois aussi, avec des visées clairement factieuses, rappelant des époques de sédition que nous pensions révolues. Nous ne cesserons de les condamner de toutes nos forces. Monsieur le Premier ministre, à l'évidence, votre Gouvernement a le devoir de résoudre une situation dont les gouvernements successifs, depuis plusieurs décennies, portent chacun une responsabilité. Nous mesurons la difficulté de votre tâche. Nul, parmi les membres du RDSE, ne souhaite votre échec, car les conséquences pour notre pays, son avenir, celui de nos enfants, seraient dramatiques. Nous nous réjouissons donc que cette colère ait pu être transformée en mots partout dans le pays, sous la forme de conférences citoyennes ou d'agoras plus spontanées et moins formalisées. Nous saluons la réussite d'un exercice complexe. La confrontation apaisée des idées est inhérente à la démocratie, puisque c'est aussi de ce concept que procède le Parlement. Pour notre part, nous sommes convaincus qu'aucune méthode n'était parfaite pour organiser ce grand débat. Les biais méthodologiques ne peuvent être éliminés d'un exercice aussi inédit dans son ampleur. La critique est un mal nécessaire et inévitable. Les quelque deux millions de contributions enregistrées sont pour nous un échantillonnage de l'état d'une certaine partie de l'opinion, celle qui s'est mobilisée. Pour autant, nous n'avons finalement rien appris que nous ne sachions déjà. Exactement ! En particulier pour des élus, comme nous qui avons été élus locaux, qui ont l'expérience de l'empathie et de l'écoute. De ces trois mois de débats, il ressort, dans les grandes lignes, de fortes demandes tendant à une fiscalité plus juste et plus lisible ; à une transition écologique moins punitive, mais adaptée à chaque territoire à une démocratie plus transparente, plus inclusive ; à des services publics mieux répartis, pour renforcer la cohésion des territoires. Monsieur le Premier ministre, le plus dur est à venir, vous le savez Tous ces échanges suscitent de l'impatience. Il est maintenant l'heure de les concrétiser par des décisions politiques, pour le court terme et pour le long terme, afin que notre pays retrouve le chemin de la fierté et de l'harmonie. Mais comment répondre à des demandes multiples, parfois incohérentes entre elles ? On ne peut pas réclamer simultanément la baisse des impôts et davantage de services publics ! Très bien ! On ne peut pas demander davantage à l'impôt et moins au contribuable. On ne peut pas promettre de réduire le poids de la fiscalité sans parler de notre politique de redistribution, un ferment de notre modèle social ! Comment ne pas surajouter de la déception aux espoirs nés ? Vous l'avez dit vous-même : « Hésiter serait pire qu'une erreur, ce serait une faute. Tout conservatisme, toute frilosité seraient à mes yeux impardonnables. » Nous voulons donc vous prendre au mot, dans l'attente évidemment des prochaines annonces du Président de la République. Ne rien faire serait bien sûr une faute. Mais continuer comme avant serait encore pire Nos concitoyens l'ont clairement dit, ils ne veulent plus d'un pouvoir vertical et déconnecté, qui fait fi des corps intermédiaires. Ils souhaitent, au contraire, que leur voix porte, au-delà des échéances électorales, ce qui n'est pas incompatible avec notre démocratie représentative. Monsieur le Premier ministre, vous nous trouverez donc à vos côtés lorsqu'il s'agira de réintroduire partout les « services publics de contact »- pour reprendre votre expression -, c'est-à-dire qui privilégient le contact humain plutôt que la chimère de la dématérialisation, de réduire les fractures territoriales, notamment en rapprochant les métropoles et les territoires périphériques, de construire une transition écologique responsable, durable et non punitive, de créer les conditions d'une meilleure répartition des richesses, par la dignité du travail. Ces combats, le groupe du RDSE les porte depuis très longtemps. Nous n'avons en tout cas jamais dévié de nos principes, dès lors que l'urgence est d'empêcher certains territoires de mourir, littéralement. Vous connaissez nos initiatives en matière de désenclavement, d'égal accès aux services publics, aux soins et au numérique, ou de développement économique des territoires. Notre engagement est constant, car nous estimons que redonner de la dignité à ceux qui se sentent oubliés exige des mesures simples, pragmatiques, adaptées au quotidien. Aussi brillante et utile soit-elle, notre technocratie n'aura jamais le ressenti du terrain des élus de proximité que nous sommes ! Monsieur le Premier ministre, l'heure est à l'action. Toutes les bonnes volontés doivent se mobiliser avec un seul objectif : mettre à jour notre logiciel démocratique, dans le respect de nos principes républicains. Pour cela, les institutions de notre démocratie représentative vont maintenant exercer leurs missions, à savoir débattre, confronter les idées, faire des propositions et voter, ce qui est le propre d'une démocratie mature. Le Sénat continuera, j'en suis sûr, de faire entendre son pluralisme et sa singularité. Mon groupe, dans toutes ses expressions et sa diversité, y prendra naturellement, avec beaucoup de détermination,

groupe. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, je dois avouer que, au début, à l'annonce du grand débat, j'étais extrêmement perplexe, j'avais un certain nombre de doutes.

la démocratie du hasard ne peut pas remplacer la véritable démocratie ! J'attends, monsieur le Premier ministre, les propositions que va nous faire le Président de la République. Je les attends avec intérêt.

la République est fragile, on vient de s'en apercevoir. Comment quelques milliers de casseurs ont-ils pu saccager, samedi après samedi, des quartiers entiers de Paris, Toulouse, Bordeaux, allant jusqu'à saccager la tombe du Soldat inconnu ? Comment quelques milliers d'individus ont-ils pu bafouer une démocratie ancienne de 67 millions d'habitants ? Comment en sommes-nous arrivés à une inversion des valeurs qui voit la violence des manifestants régulièrement « comprise » et les forces de l'ordre systématiquement soupçonnées ? Ces questions ne figuraient pas à l'agenda du grand débat. Elles auraient pourtant constitué un point d'entrée stimulant pour saisir les maux de notre société. Ce grand débat ausculte un malaise, une colère venus de loin et du plus profond de nos territoires, dont le mouvement initial des « gilets jaunes » a été un impitoyable et juste révélateur. Aura-t-il eu une utilité s'il n'aborde pas aussi quelques questions mises sous le tapis depuis cinquante ans ? Par exemple, sur le respect dû à autrui, sur le sens de l'autorité, sur la prééminence de l'intérêt général ? Servira-t-il à quelque chose si la montée de la violence, sous toutes ses formes, n'est pas traitée ? Servira-t-il à quelque chose si le délitement du civisme et de la responsabilité individuelle n'est pas abordé ? Servira-t-il à quelque chose si la norme, le traité et le juge asphyxient la volonté politique ? Le Gouvernement nous dit que le grand débat est un succès, c'est vrai. Permettez-moi d'apporter toutefois quelques nuances. Les manifestants sincères de novembre ont rarement rejoint les salles de réunion. Quant aux manifestants « professionnels », ils n'ont évidemment pas joué le jeu d'un dialogue qu'ils méprisent. Ils nous le disent chaque samedi, pavé à la main ! Il faut naturellement remercier les nombreux Français qui ont fait la démarche d'échanger et de s'écouter. remercier à mon tour les milliers d'élus locaux, les maires qui ont organisé et animé ces réunions, ce sont les grands gagnants du débat, ils ont enfin été réhabilités. Ils ont rendu possible une photographie de l'opinion à un moment important. Cette photographie est cependant partielle. Partielle, car ces contributeurs ne constituent pas un échantillon représentatif. Toutes les classes d'âge, toutes les classes sociales, tous les types de territoires n'étaient pas également présents dans les salles de réunion ou dans les contributions, tant s'en faut. Il en résulte ainsi des idées parfois innovantes, stimulantes. Néanmoins, elles n'ont pas la légitimité à s'imposer en tant qu'opinions dominantes. Des Français se sont exprimés. Ils ne sont pas tous les Français, ils ne sont pas la France, comme vient de le dire Claude Malhuret avec talent. La légitimité démocratique est à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, ici au Sénat, et dans les mairies. Elle peut être dans des référendums ou des consultations populaires plus nombreux et plus ouverts que nous appelons de nos voeux, elle n'est nulle part ailleurs. Le droit de pétition, oui, le mandat impératif, non La photographie du grand débat est également partiale. Les sujets qui avaient été sélectionnés sont fondamentaux. Le Gouvernement a eu raison de provoquer une réflexion collective autour d'eux. Mais comment justifier que d'autres n'aient pas été traités ? Quasiment aucune question sur notre rapport à l'Europe, sur l'innovation, sur l'impact des nouvelles technologies, sur l'immigration et l'intégration, sur le fonctionnement de la justice, sur la sécurité, sur le terrorisme. Ces sujets ne sont pas moins importants. Je note d'ailleurs qu'il ressort de la consultation les préoccupations que les sénateurs, ancrés dans la terre fertile de leurs départements, signalaient de longue date, l'accès aux soins, à la formation, à internet, à la mobilité. Pour autant, les élites vilipendées, auxquelles certains Français nous associent, auraient mauvaise grâce de pointer les seules lacunes ou contradictions. En effet, si un seul élément ressort du débat, c'est notre perte de crédibilité, notre indispensable introspection et le besoin d'agir différemment. À ce titre, deux aspects de la crise sociale de l'automne restent cruciaux : d'abord, les sentiments de mépris et d'abandon, particulièrement ressentis dans les villes moyennes et nos campagnes ; ensuite, le sentiment d'injustice à l'égard des efforts à fournir pour faire avancer le lourd char de l'État, conduisant nos concitoyens Le manque de considération, voilà l'un des maux de notre époque, vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre. Il est façonné par la conviction que les élites parisiennes prennent des décisions déconnectées. Notre groupe est historiquement convaincu des bienfaits de la logique de subsidiarité. Cela s'appelle décentraliser et différencier. Décentraliser, parce que plus la chaîne d'analyse, de décision et d'évaluation est courte, plus la probabilité que l'action publique soit appropriée est élevée. C'est vrai ! Nous appelons ainsi à un acte III de la décentralisation et à un terme, enfin, aux doublons insupportables. à une « clarification » et à de « vrais choix », comme le dirait le Président de la République. Mais décentraliser ou déconcentrer ne sont plus suffisants, il faut ouvrir des espaces, des espaces de différenciation. Il ne suffit plus de dire que telle collectivité gérerait mieux que l'État telle politique publique, il faut lui donner la capacité d'adapter cette politique à son territoire. On ne structure pas nécessairement de la même façon les dispositifs d'insertion dans la Creuse et dans le Val-de-Marne. Nous sommes nombreux à être ouverts à ce bon sens. Si ce n'est que nous allons vite ouvrir un débat très français : sera-t-il juste que l'allocation de parent isolé soit de 20 euros moins élevée en Lozère qu'en Essonne ? Sera-t-il juste qu'un ascenseur soit obligatoire dans les immeubles de trois étages en région parisienne quand il ne le sera pas en province ? Nous devons pouvoir assumer ces disparités, dès lors qu'elles sont encadrées par le législateur, avec le souci de l'unité républicaine. Très bien ! Pour notre part, nous faisons confiance aux élus locaux et nous appuierons cette orientation. Mais renforcer les marges d'action des élus locaux suppose que les citoyens puissent mesurer l'efficacité de leurs actions. L'article 72 de notre Constitution doit ainsi être précisé. Les élus doivent s'appuyer sur une réelle autonomie financière. Les citoyens doivent être confrontés à une fiscalité redevenue simple et lisible. L'injustice est le maître mot depuis décembre. Il ne l'était pas en novembre, lorsqu'il s'agissait de dénoncer de nouvelles taxes. Le logiciel des quarante dernières années s'est remis en marche et a souvent transformé le débat sur le trop-plein d'imposition en débat sur l'injustice fiscale, permettant ainsi de ne pas s'interroger sur l'efficacité de la dépense publique à la française, pourtant triste championne du monde. Dans notre pays passionné d'égalité, le sentiment d'injustice est omniprésent et facile à alimenter. Cela ne doit pas empêcher de dénoncer les incohérences qui minent notre contrat social. Il est évident que certaines entreprises ne paient pas leur dû. Il est évident que certaines optimisations fiscales n'ont guère de légitimité. Il est évident que la fraude sociale est trop importante. Il est évident que la confusion règne entre assistance et assurance. Il est évident que la lenteur de la justice alimente le sentiment d'impunité. Se focaliser sur les seules inégalités est une voie sans issue. Notre énergie gagnerait à se concentrer simultanément sur deux dimensions, créer de la richesse et faire mieux fonctionner les services publics. En créant de la richesse, nous nous dotons de la capacité à réformer dans le sens d'une plus grande justice. Dans notre pays attaché aux positions acquises, seules des évolutions au temps long avec des sorties par le haut sont réalistes. Elles ont un coût. Seules des ressources nouvelles peuvent les financer. Pour cela, il faut de la croissance. Le moment venu, chacun devra faire des propositions précises. Notre groupe a ainsi d'ores et déjà apporté sa contribution en matière fiscale- notamment par la voix de Vincent Delahaye -, contribution qui répond d'ailleurs à l'exaspération des Français. Des services publics ambitieux sont, par ailleurs, le meilleur outil de lutte contre les inégalités. Savoir lire et compter dès l'âge de six ans, être protégé des délinquants où que l'on habite, être vite et bien soigné à l'hôpital sont les meilleurs services à rendre aux plus démunis. Encore faut-il que ces services soient performants. Nous demandons ainsi au Gouvernement de se concentrer sur la poursuite de réformes maintes fois anéanties par le conservatisme. Cela sera beaucoup plus efficace ! Monsieur le Premier ministre, les conditions de l'élection présidentielle nous ont privés d'un réel débat. Ce débat, nous venons de l'avoir parce qu'un débat vaut mieux qu'une émeute, c'est évident Mais un débat n'est qu'un outil d'aide à la décision. Après la restitution vient le moment des choix. Les institutions républicaines doivent reprendre leur place. La rivière doit rentrer dans son lit. Il appartient aujourd'hui au Président de la République et à votre gouvernement d'exprimer ses conclusions.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des orateurs qui se sont succédé à cette tribune pour la qualité et la mesure de leurs propos. Les critiques peuvent être vives, mais il me paraît que nous avons eu un échange de qualité. Je le dis, parce que j'ai connu non pas des assemblées, mais des moments où les débats étaient moins que celui-ci et je voulais en remercier le Sénat. J'ai peu de choses à ajouter, mesdames, messieurs les sénateurs, à ce qu'a dit avec un immense talent et une très grande lucidité le président Malhuret.Je voudrais remercier le président Patriat pour son extraordinaire soutien. C'est vrai que J'ai appris à mesurer que, lorsque les temps sont difficiles, avoir des soutiens fidèles est quelque chose d'utile Je veux le dire, je me retrouve dans beaucoup des éléments qui viennent d'être développés par le président Marseille. Permettez-moi d'insister sur quelques mots évoqués par plusieurs des orateurs,

que les voies d'accès au grand débat soient les plus diversifiées possible, de façon à réduire, globalement, les biais. Je crois que c'est ce que nous ont dit les garants

manifester avec pour seule revendication la violence. Il me semble que nous devons à tout le moins assumer le fait que nos concitoyens ont voulu se saisir d'un espace démocratique pour dire ce qu'ils souhaitaient. Cela a été, de ce point de vue- je le dis et je l'assume -, un grand succès. Je suis Je suis pleinement en accord avec le président Retailleau quand il déclare son attachement aux institutions de la V République. J'y suis tout autant attaché que lui.

qu'il est la clé de voûte des institutions ; il lui reviendra donc d'annoncer les décisions prises à l'issue de ce grand débat. Cela suscite de très grandes attentes

par le travail et que l'épanouissement individuel passe lui aussi par le travail. Vous avez rappelé, monsieur le président Retailleau, que j'ai eu l'honneur d'être maire d'une grande et belle commune, celle du Havre. Je vous en remercie : je ne l'ai pas oublié du tout, et je ne crois pas que je pourrais un jour

Je me souviens de l'annonce, une semaine après les élections municipales de 2014, d'une diminution massive et régulière des subventions aux collectivités territoriales. Je m'en souviens parfaitement : ce n'était pas anxiogène,

ce que nous savons tous, à savoir le caractère contradictoire d'un certain nombre d'expressions des Français. Le consensus peut intervenir sur des objectifs généraux, généraux, il peut intervenir sur des sujets précis, mais notre pays n'est pas un pays de consensus : c'est un pays de débats, c'est un pays d'oppositions. Au fond, c'est ainsi qu'on l'aime Ce ne serait pas une démocratie, ce ne serait certainement pas notre République s'il venait à changer. Il serait intéressant- vous l'avez dit, monsieur le président Requier -de faire en sorte que, sur les éléments de consensus,

elles sont souvent utiles, mais je ne crois pas que le renvoi à une grande conférence soit de nature à répondre, à lui seul, aux exigences et aux demandes que les Français ont exprimées pendant le grand débat. J'ai le souvenir, là encore, de grandes conférences

Il est assez largement contraire aux exigences médiatiques de notre époque. Lorsque nous travaillerons à l'élaboration de compromis démocratiques, nous le ferons sous la pression et face à l'insatisfaction de ceux qui nous observent. Nous le savons tous ici. Pourtant, je suis convaincu que nous devrons construire ces compromis et travailler avec les corps intermédiaires pour atteindre les objectifs qui ont été

Je voudrais aussi revenir sur la question de la conjugaison entre la démocratie représentative et d'autres formes de démocratie qui sont nécessaires,

Nous aurons l'occasion d'en redire un mot, madame la présidente Assassi, notamment à propos de l'initiative qui a été prise récemment en matière de référendum d'initiative partagée. Le texte

Les Français ont manifesté leur mécontentement et leurs inquiétudes. Aujourd'hui, notre modèle social, qui était la base de notre pacte national, est attaqué de toutes parts. Son financement est déséquilibré : certains paient toujours plus, car la base contributive diminue sans cesse du fait du vieillissement de la population et du chômage. Pourtant, les besoins n'ont jamais été aussi forts. Les attentes exprimées lors du grand débat national sont importantes. La paupérisation de ceux qui ont travaillé toute leur vie n'est ni digne ni tolérable. La régulation des soins par la pénurie ne l'est pas non plus. Lorsqu'on évoque les grands sujets que sont la dépendance ou le handicap, le financement est renvoyé à plus tard. Madame la ministre des solidarités et de la santé, pensez-vous toujours pouvoir faire en sorte que les Français puissent bénéficier d'un haut niveau de solidarité ? Les premières mesures portées par le Gouvernement concernant les retraités et la santé ne vont pas forcément dans ce sens. Or le Gouvernement ne sortira de la crise que si elle est l'occasion, pour lui, de faire oeuvre de vérité. Cela passe par la valeur travail, et non par l'augmentation de la dette et des déficits.

et nous ne souhaitons en aucun cas le dégrader ; nous avons même l'ambition de l'améliorer encore, par la couverture d'un nouveau risque dont nous avons largement parlé et qui a émergé du grand débat : celui du grand âge, de la perte d'autonomie et de la dépendance. les problèmes de nos Ehpad et des professionnels qui y travaillent. Nous avons le devoir d'affronter en face la réalité d'une population qui vieillit et qui va avoir des besoins supplémentaires.

Le mouvement des « gilets jaunes » traduit une fracture territoriale liée aux conséquences de la numérisation de l'économie. Celle-ci favorise les métropoles, lesquelles ont du mal à loger les travailleurs qu'elles attirent, au détriment d'autres territoires qui souffrent. Le numérique, c'est ce que nous avons tous dans nos poches,

pétitions, appels à manifester de façon masquée, tout cela représente une révolution qui a, elle aussi, rendu possible le mouvement des « gilets jaunes » tel qu'il s'est déroulé. Alors, comment mener des politiques publiques dans un monde numérique ?

des règles qui peuvent être liées à la manipulation de l'information. Il faut faire en sorte que les règles qui s'appliquent dans la vie de tous les jours s'appliquent aussi sur internet. Ensuite, pour qu'internet soit un outil au service de la démocratie, encore faut-il que les gens y aient faut donc réduire la fracture numérique, qui s'est creusée depuis quelques années dans notre pays. C'est notamment la mission que se sont assignée Jacqueline Gourault et Julien Denormandie, de manière à ce que tous nos territoires puissent bénéficier d'un bon débit. d'organiser la présence de l'État dans les territoires afin de donner accès à ces outils numériques, de former les gens qui ne savent aujourd'hui se servir ni d'un clavier ni d'une souris ; ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne peut le penser. Ainsi,,

Surtout, ne nous dites pas que l'IFI que vous proposez fera oeuvre de justice sociale ! En effet, 80 % du patrimoine des ménages les plus aisés est composé de capital mobilier. Les richesses d'aujourd'hui, ce ne sont plus l'usine à papa et les grands domaines ; ce sont des sommes immenses, des actions, des obligations volatiles qui s'accumulent dans les poches de quelques-uns, particulièrement à l'heure du numérique. Monsieur le Premier ministre, allez-vous écouter les Français et enfin rétablir l'ISF ? que candidat, votre ami Emmanuel Macron déclarait : « La TVA, c'est injuste. » Pour ma part, je pense à Corinne, ma concitoyenne d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Elle me demande de vous interpeller, parce que des produits aussi importants que le savon, le dentifrice ou les pâtes sont trop chers. C'est aussi le cas des protections hygiéniques, taxées à 5,5 %. Les femmes sont contraintes à un nombre de dépenses considérablement plus élevé vivent avec 20 % de salaire en moins ! Monsieur le Premier ministre, fixer à 0 % le taux de la TVA sur les produits de première nécessité n'est pas seulement, pour reprendre votre propos, intellectuellement possible ; c'est urgent Que répondez-vous à Corinne et, à travers elle, à l'ensemble des citoyens de ce pays ? Il faut conclure ! Comptez-vous donner un calendrier pour la réalisation de cette mesure, demande incessante de nos concitoyens

Ce que nos concitoyens demandent, c'est d'être en mesure de vivre décemment de leur travail, c'est de ne pas avoir à compter chaque euro lorsqu'ils remplissent leur caddie, c'est de ne pas être tous les mois systématiquement à découvert, c'est de ne pas s'endetter pour payer des factures liées au logement et à l'électricité, c'est de ne pas avoir à renoncer Les inégalités sociales se creusent et sont le reflet d'un partage des richesses profondément injuste. Les mobilisations citoyennes que nous connaissons depuis plusieurs mois parlent d'elles-mêmes. La réponse que le Gouvernement doit apporter à ces mouvements sociaux inédits consiste à résoudre l'équation

par les dépenses liées au logement ? Les locataires modestes sont les premières victimes des coupes budgétaires sur les allocations logement et de la hausse du prix de l'électricité qui s'annonce. Ils subissent une double peine : l'impossibilité de s'acquitter des dépenses courantes et une assignation à des logements moins-disants et plus énergivores. 7,4 millions de foyers vivent dans des logements mal isolés, ils subissent les conséquences d'un marché insuffisamment réglementé et supportent des dépenses qui devraient être à la charge du bailleur. La justice consiste à anticiper les problèmes et non pas à panser les plaies d'une société encore trop inégalitaire. Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et venir en aide aux familles les plus en difficulté ?

Karoutchi. Depuis la royauté, la France s'enorgueillit d'accorder l'asile à tous les persécutés. Depuis la République, elle conduit une politique d'assimilation, puis d'intégration, pour que les nouveaux arrivants participent à l'unité de la Nation et s'approprient les principes de la République. ces deux modèles sont à bout de souffle. Le droit d'asile est détourné par des filières d'immigration économique ou sanitaire et l'intégration des nouveaux arrivants se heurte au problème

Monsieur le Premier ministre, défendre la République, c'est aussi défendre l'unité de la Nation et cette vision de la société française. Allez-vous oui ou non mettre en place une politique ferme, mais juste, qui intègre sans faire courir de risques à la République ?

Depuis le mois de novembre dernier, le mouvement des « gilets jaunes » a rendu visible la défiance que nos concitoyens nourrissent à l'égard de nos mécanismes démocratiques. Animés par le sentiment d'être déconnectés de l'élaboration des politiques publiques, ils s'insurgent aux fins d'être plus régulièrement consultés et intégrés dans le des décisions. Dans le grand débat national, le Gouvernement a confié à près de 700 médiateurs, facilitateurs de parole, la lourde tâche de transformer une contestation violente en une concertation constructive, la responsabilité d'animer et de réguler au plus près du terrain ces participations de citoyens aspirant à devenir bien plus que de simples administrés. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Nous disposons d'outils originaux qui ne demandent qu'à être développés,

témoigne de la volonté de revivifier l'expression de la citoyenneté. Cela peut se faire de mille et une manières, par exemple en associant des citoyens

faut engager un travail pour instiller des éléments de démocratie participative dans notre vie politique et dans notre vie démocratique. Cela peut prendre différentes formes. Celle que vous proposez en est une, même si je ne sais pas si cela doit être imposé

acceptée et efficace, quelle est la vision du Gouvernement sur l'avenir de la fiscalité écologique, sans laquelle il ne peut y avoir de véritable transition écologique ? La parole

il est temps de passer du débat aux actes. L'inscription dans les programmes scolaires dès le primaire de cours de sensibilisation à la transition énergétique serait un début. Alors que l'urgence climatique et environnementale nous commande de revoir entièrement notre modèle énergétique, toute l'attention est focalisée sur la production. Or un problème majeur semble avoir été sous-estimé, celui de la refonte énergétique du parc de logements français, notamment du parc ancien. L'un des moyens les plus efficaces est de diminuer les consommations énergétiques à la source, c'est-à-dire au sein même des foyers. Environ 4 milliards d'euros sont mobilisés chaque année pour l'habitat sous des formes multiples. Ces fonds publics et privés sont censés aider à la rénovation de 550 000 logements privés et autour de 100 000 maisons et appartements. Ces chiffres figuraient dans la loi de 2015, avec l'ambition de rendre le parc immobilier vertueux d'ici à 2050, avec une éradication des passoires thermiques d'ici à 2025. Malheureusement, du retard a été pris, et il faudrait presque aller deux fois plus vite. Et que dire des ménages

quelles actions concrètes le Gouvernement compte-t-il engager pour simplifier et rendre plus lisibles les outils et aides actuels en matière de rénovation énergétique dans le logement et ainsi les rendre réellement incitatifs et attractifs pour tous les ménages ?

Il y a concrètement des gains de pouvoir d'achat possibles par la transformation écologique, notamment celle de nos logements, qui permet notamment de réduire les factures de chauffage.

les soins de ville, quant à eux, souffrent d'une désertification médicale, le secteur libéral ayant été affaibli sans alternative durable. Nous partageons également tous l'objectif que les patients puissent tous avoir un médecin traitant, accéder à un médecin spécialiste dans des délais raisonnables et être accueillis dans des hôpitaux mieux organisés avec des personnels

Quant aux communautés professionnelles territoriales de santé, elles sont un modèle d'organisation uniforme. C'est un modèle centralisateur, qui ne correspond en rien à la diversité de nos territoires. Madame la ministre, pourquoi le Gouvernement s'obstine-t-il à à poursuivre des mesures qui augmentent le temps administratif des médecins et ne libèrent pas de temps médical

Dans un récent entretien à, le ministre Sébastien Lecornu a mis en avant cette proposition, qui permettrait notamment de réaliser des économies, en diminuant le nombre d'élus sans remettre en cause l'existence du conseil régional et du conseil départemental, à la différence de ce qui a été imaginé en son temps par le gouvernement Fillon. Je partage cette proposition. Chacun sait bien que le conseiller régional n'a jamais connu la même légitimité que le conseiller départemental, qui est beaucoup plus reconnu par les acteurs locaux et plus engagé localement sur un territoire bien identifié.

il faudrait veiller à préserver la parité, à éviter une explosion de la taille des assemblées régionales, à affirmer l'ancrage local de tous les élus locaux, ... Il faut conclure ! ... et ce dans le respect de la règle d'égalité pour représenter un territoire dans une assemblée, qu'a posée le Conseil constitutionnel.

Notre devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » est remplacée progressivement par « libéralisation, concurrence, privatisation ». Pourtant, les « gilets jaunes », comme une majorité de Français, refusent qu'on confie au privé nos biens communs. Les libéraux avaient promis que la concurrence conduirait à une baisse des prix et à un meilleur service. Or les Français observent chaque jour que les prix augmentent pour les usagers devenus des clients- 6 % pour l'électricité l'été prochain -, que les salariés sont la variable d'ajustement et que les profits s'envolent au bénéfice des actionnaires. Les Français sont majoritairement contre la privatisation des barrages hydroélectriques et pour une renationalisation des autoroutes, ce qu'a défendu notre groupe le mois dernier et que vous avez refusé. Français s'opposent à la future privatisation d'Aéroports de Paris, monopole naturel au regard de ses 100 millions de passagers par an. C'est une question de souveraineté nationale, de sécurité, d'aménagement du territoire, mais aussi une question économique, sociale et environnementale. L'an dernier, ADP a versé 180 millions d'euros à l'État en tant qu'actionnaire. Nous refusons que cet argent aille engraisser les actionnaires de Vinci, car cet argent serait plus utile à nos hôpitaux et nos écoles. Pourquoi vous entêtez-vous à privatiser ADP au profit des riches, plutôt que de défendre nos biens communs qui sont le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas ? Si vous êtes si sûr de vous,

Grâce au travail qui a été accompli au Parlement- au Sénat et à l'Assemblée nationale -, nous avons renforcé les garanties sur les tarifs, l'environnement, la récupération du foncier, la manière dont l'entreprise sera gérée, les investissements nécessaires et le cahier des charges, qui vous a été fourni.

Vous avez pris l'initiative de demander un référendum d'initiative partagée, dans un attelage étrange qui est peut-être la première étape d'un programme commun entre Les Républicains et le parti socialiste.

Je constate d'ailleurs que, dans leur grande sagesse, ni le président du groupe Les Républicains au Sénat ni le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale ne se sont associés à cette initiative, sans doute parce qu'ils la trouvaient surprenante, voire déplacée. Ils y viendront ! Ce que je constate, Ce que je constate, monsieur Gay, c'est que vous affaiblissez la démocratie représentative en contestant les dizaines d'heures de travail de nos représentants- sénateurs et députés -sur la privatisation d'ADP et, avant même que le projet de loi ne soit voté,

Le Gouvernement a lancé ce grand débat en posant la question du niveau des prélèvements obligatoires. Or nous pensons que la question qui est posée par les Français, c'est celle de la justice fiscale. Ce n'est pas la même chose Les principales raisons des contestations qui s'expriment vivement depuis novembre proviennent de l'accroissement des inégalités, devenues insupportables après les premières décisions budgétaires que vous avez prises dès 2017. L'abaissement des mécanismes de redistribution est multiforme : baisse des APL, réduction des emplois aidés, hausse de la CSG pour tous les retraités, plan Pauvreté en deçà des attentes. Vos choix ont ainsi abouti à une remise en cause de notre pacte social dans des proportions jamais vues sous la V République. La fin de l'ISF a eu des effets désastreux en matière d'acceptabilité de l'impôt. Cette suppression, couplée à la mise en place de la, a permis à chacun des

à notre Président, est dans les faits clairement déséquilibrée en faveur des contribuables les plus fortunés. Nous nous interrogeons sur vos ambitions en matière de lutte contre les inégalités fiscales. Si vous continuez à nous dire, comme M. le ministre de l'économie, que, pour lutter contre l'injustice fiscale, il faut réduire l'impôt, c'est pour nous un aveu clair : vous refusez de traiter la question essentielle de l'équité contributive

nous en avons supprimé -, puis la TVA. La question se pose de son équité et de son acceptabilité, selon ses moyens contributifs. Nous n'avons pas, dans un premier temps, posé la question de la TVA. D'autres la posent, y compris d'ailleurs dans votre famille politique désormais.

Qui regarde les comptes publics sait que c'est faux ! Instaurer une taxe carbone et baisser les budgets consacrés à l'environnement ne trompent pas nos concitoyens. Annoncer que vous baissez les impôts en comptabilisant ceux que vous aviez prévus et auxquels vous renoncez, c'est incroyable ! Ce que nos compatriotes attendent maintenant, ce sont des faits des chiffres clairs de baisses d'impôts. Alors, allez-vous supprimer l'augmentation de la CSG pour tous les retraités ? Quels impôts va-t-on voir enfin baisser ? Et quand ? Quel niveau de prélèvements obligatoires vous fixez-vous comme objectif ? Plus votre réponse sera précise, plus elle sera convaincante. Les Français nous regardent

Notre philosophie, pour vous répondre sur le type d'impôts que nous souhaitons baisser, c'est d'aider d'abord ceux qui travaillent. Je pense que vous serez d'accord avec nous sur ce point, comme un bon nombre de vos collègues sur les travées du Sénat : il faut aider principalement ceux qui travaillent pour que le travail paie davantage et que tous ceux qui ont un emploi aient le sentiment qu'ils peuvent en vivre

plus efficacement aux réalités des territoires. Ce souhait, nous ne pouvons que le partager. Il est temps de redonner de la cohérence à une organisation territoriale profondément abîmée et déstructurée par les réformes antérieures, notamment par la loi NOTRe. Il est nécessaire de restaurer une meilleure lisibilité de la carte territoriale, mais également de donner aux collectivités les moyens de leurs compétences. En parallèle, l'État doit assumer son rôle dans nos territoires, notamment dans les plus fragiles d'entre eux, où les habitants considèrent souvent qu'ils sont traités comme des citoyens de seconde zone. C'est la raison pour laquelle je pense en effet que les préfets doivent voir leur pouvoir de décision renforcé et surtout- surtout ! -adapté aux territoires dont ils ont la charge. Il est également nécessaire de donner à ces territoires, qui font la fierté de notre pays, les moyens de leur développement économique. Madame la ministre de la cohésion des territoires, comptez-vous lancer le chantier d'une grande réforme territoriale ?

conserver une organisation territoriale de l'État forte. Nous savons combien les élus et la population sont attachés à la présence des services de l'État sur le territoire.

Dans les petites communes, au-delà de la fermeture sans négociation des services publics- écoles, hôpitaux, agences du trésor public, bureaux de poste, etc. -, il existe sur le plan financier une injustice aussi fondamentale qu'insupportable

Et n'exercerait-elle pas aujourd'hui ces compétences transversales ? Quels que soient les montants de la DSU, de la DSR et des péréquations, l'État peut-il concevoir qu'un Français vaille deux fois plus à un endroit qu'à un autre ? Dès son élection, le Président de la République a annoncé la suppression de la taxe d'habitation au motif qu'elle était un impôt injuste. Monsieur le Premier ministre, la dotation de base de la DGF est-elle juste ? Allez-vous rendre justice au monde rural et aux petites communes ? La parole est à M. le ministre de l'action et des comptes publics. Madame

qui relèvent de la politique de la ville, et sur les intercommunalités, en plein développement. Or je constate que tous ceux qui ont essayé de réformer la DGF et toutes les dotations depuis le gouvernement Barre ont échoué. Il appartient sans doute à la Haute Assemblée de s'y intéresser particulièrement- je sais que vous le faites -, mais aussi aux élus locaux et au Comité des finances locales.

11 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, c'est positif. Il faut faire évoluer l'organisation de l'État et des services publics pour plus d'efficacité et un meilleur rééquilibrage. Il faut renforcer les dotations aux communes, soutenir l'aménagement des centres-bourgs, développer internet et la téléphonie mobile, restructurer le réseau ferroviaire et les lignes Intercités secondaires, maintenir les écoles, les gendarmeries, les sapeurs-pompiers volontaires, car ils sont indispensables, développer l'emploi par les entreprises par l'intermédiaire d'un préfet développeur, grâce à des zones franches et des ZRR efficaces. De plus, il faut

mes questions : comment, dans ces territoires hyper-ruraux, adapter le rôle de l'État pour le rendre plus efficace, pour l'emploi et le service public, pour y maintenir la vie ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour supprimer les zones blanches en matière de santé et maintenir les centres de secours ?

de nos communes, il est un échec dont vous portez l'entière paternité, c'est à l'évidence celui de la Conférence nationale des territoires. Cette conférence, dont le Président de la République lui-même attendait des propositions concrètes, n'a pas été capable de corriger ce que vous appelez vous-mêmes « les irritants » de la loi NOTRe. Il a fallu que le Sénat

de retrouver la voie de l'espérance. Au cours du grand débat national, le Président de la République a avancé un nombre incroyable de pistes. J'ai envie de dire : finies les paroles, place aux actes ! Il est temps pour vous de conjuguer le « dire » et le « faire » et de reprendre les propositions du Sénat. Il n'y a, comme disait Churchill, aucun mal à changer d'avis, pourvu que ce soit dans le bon sens ! La parole

pour celles et ceux qui adhèrent à un régime d'assurance maladie dans un pays membre de l'espace économique européen et en Suisse. Ils

de traités européens, qui garantissent un certain nombre de droits. Pour les résidents européens, ces droits sont la libre circulation des personnes et des marchandises dans l'Union. Il n'y a rien d'anormal à ce que les traités créent des régimes juridiques différents pour les résidents européens et extra-européens. En l'occurrence, la différence de traitement que vous mentionnez trouve une traduction en matière sociale avec l'exonération de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital, qui ne concerne en effet que les résidents de l'Union européenne. Il faut toutefois préciser que, en l'espèce, c'est non pas le critère de résidence qui joue, mais celui de l'affiliation. L'assujettissement aux cotisations et aux contributions sociales dépend du système social d'affiliation. Toutes les personnes affiliées au système français de sécurité sociale sont soumises aux mêmes règles. Inversement, la coopération européenne et la coordination en matière de sécurité sociale imposent que les affiliés aux autres systèmes sociaux européens puissent n'être soumis qu'aux règles de ces autres systèmes. Ces garanties existent entre systèmes européens en raison d'objectifs convergents et comme contrepartie à la coordination qui existe entre eux. En dehors de l'Union européenne, il est normal que le principe de territorialité s'applique en l'absence de coordination entre les systèmes sociaux, sauf lorsqu'il existe des conventions spécifiques.

rien de surprenant à cela. Nos concitoyens vivent en effet douloureusement la destruction conjuguée des deux piliers de notre système d'accès aux soins que sont la médecine de ville- les déserts médicaux progressent de manière très inquiétante -et l'hôpital public, lequel est aujourd'hui à l'os et ne tient plus que grâce à l'exceptionnel engagement de ses personnels. Personne n'acceptera que l'examen de la loi Santé se poursuive comme si de rien n'était. Personne n'acceptera qu'après avoir fait les questions de ce grand débat, vous en fassiez aussi les réponses Le conventionnement sélectif des médecins doit être décidé pour commencer à corriger au plus vite la démographie médicale en dissuadant de nouvelles implantations dans des zones surdotées. Des propositions ont été travaillées ici même en ce sens, elles peuvent rapidement voir le jour. Le système libéral étant incapable de se réguler, il est nécessaire que la puissance publique intervienne pour développer les unités employant des médecins salariés. Il faut donc aussi soutenir les centres de santé, portés notamment par les collectivités locales. Il est enfin urgent non seulement de mettre fin aux fermetures de maternités et d'hôpitaux de proximité, mais également de rouvrir un certain nombre d'entre eux. Comptez-vous prendre en compte ces propositions ?

En matière de transition écologique comme de volontarisme institutionnel, on attendait du Gouvernement des propositions plus éclatantes que le recyclage du conseiller territorial, avec ses justifications managériales d'efficacité et d'économies. Encore une incompréhension majeure sur ce que doit véritablement être la démocratie de proximité ! Recentrons-nous plutôt sur une fonction curieusement absente du grand débat : la fonction présidentielle. Je comprends bien qu'affaiblir les assemblées, cultiver l'antiparlementarisme, supprimer les contre-pouvoirs, des corps intermédiaires jusqu'aux représentants du personnel, offre un confort incomparable. C'est d'ailleurs ainsi que l'ultralibéralisme produit mécaniquement des dérives autoritaires, sous couvert de neutralité technicienne. En dépit de ce qu'on essaie de faire dire aux Français après le grand débat par un exercice de ventriloquie déconcertant de candeur, ce n'est pas ce qu'ils attendent pour la France ni d'ailleurs pour l'Europe.

Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous prendre en considération le grand débat dans le cadre d'une révision institutionnelle sans cesse reportée ? Allez-vous transformer ce qui est un projet de technocratie plébiscitaire et de domestication du Parlement en une opportunité pour rééquilibrer notre architecture institutionnelle en faveur d'une meilleure représentation des citoyens et des corps intermédiaires ? Allez-vous accepter de mettre en place de nouveaux mécanismes délibératifs ... Il faut conclure ! ... et représentatifs pour revitaliser une V République épuisée par une présidentialisation excessive ?

votre question est assez paradoxale. Le Premier ministre l'a dit, le grand débat a fait émerger des questions fortes, il a également été marqué par un certain

de le repositionner. En revanche, je vous rejoins assez aisément lorsque vous soulignez une demande d'évolution de la démocratie telle qu'elle s'exerce aujourd'hui pour y introduire, je le disais, des éléments de démocratie participative.

Ce cri correspondait à la fracture territoriale illustrée par les problèmes de mobilité, l'absence de services publics, la fiscalité, les 80 kilomètres à l'heure, le pouvoir d'achat et des revenus « inadmissiblement » bas. Dans ma commune comme ailleurs, la moyenne mensuelle des retraites agricoles est inférieure à 600 euros. La France devrait avoir honte. Cependant, le problème le plus dangereux pour la survie de la ruralité est la santé, très souvent citée dans le grand débat. Les médecins généralistes arrivent à la retraite et ne sont pas remplacés. Pour une visite chez un spécialiste, il faut attendre un an et parcourir cent kilomètres aller-retour en voiture en l'absence de transports en commun. La ruralité attirait de plus en plus de retraités lassés de la ville, mais ceux-ci ne viendront plus sur un territoire sans médecin, sans dentiste, avec la pharmacie fermée et les cabinets d'infirmiers partis. Dans ma question d'actualité du 30 octobre dernier, j'appelais l'attention sur le mouvement du 17 novembre. Bien entendu, le Gouvernement n'avait pas compris et il a été sourd à cet appel au secours. On a vu la suite ... M. de Rugy n'a d'ailleurs toujours pas compris ! Les propositions homéopathiques contenues dans la loi Santé ne changeront rien, comme tout ce qui a été fait depuis de très nombreuses années. Il convient de prendre des décisions énergiques, autoritaires et en partie coercitives pour ne pas laisser sans soins des millions de Français. Les ruraux ne veulent pas de soins palliatifs, mais des soins curatifs. La ruralité a la jaunisse, ... Votre question ! ... vous ne la soignerez pas avec un cachet d'aspirine et des belles paroles. Madame la ministre de la santé, que comptez-vous faire pour que des millions de Français puissent encore se faire soigner ? Madame la ministre de la santé,

à un médecin traitant, à des soins non programmés, à la prévention. Des organisations nouvelles vont se mettre en place dans les territoires. Nous allons doubler les maisons de santé et les centres de santé pluriprofessionnels, car c'est l'avenir de la médecine. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde aujourd'hui. La médecine en cabinet isolé est vouée à disparaître, parce qu'elle n'est plus adaptée pour soigner les pathologies chroniques. Nous allons structurer des hôpitaux de proximité qui rendront un service proximité autour de la gériatrie, de la médecine polyvalente, de plateaux techniques. Nous allons réinvestir dans ces hôpitaux. Nous allons y favoriser des consultations avancées de spécialistes,

nos concitoyens attendent du Président de la République et du Gouvernement des mesures concrètes susceptibles d'avoir une traduction effective à court terme. Dans l'esprit des Français, il s'agit essentiellement de mesures à caractère fiscal et en faveur du pouvoir d'achat. Le Premier ministre a lui-même évoqué « une immense exaspération fiscale », mais si cette exaspération porte sur le niveau global des prélèvements, elle s'adresse aussi à la répartition de l'effort fiscal. Pouvez-vous imaginer une réforme fiscale sans que celle-ci concerne aussi la TVA ? L'institution d'une TVA à taux zéro sur certains produits de première nécessité, les produits alimentaires non transformés par exemple, et l'application d'un taux réduit à une gamme plus large de produits incluant en particulier des produits d'hygiène concourant à des objectifs de santé publique sont une réponse en termes de pouvoir d'achat. Je connais les objections récurrentes du ministère de l'économie et des finances sur de telles propositions. L'argument selon lequel le différentiel de TVA serait capté par une majoration de la marge des producteurs et des distributeurs me paraît infondé, car nous sommes bien dans une économie de marché, donc concurrentielle, et cela prouverait par l'absurde que les taux intermédiaires et réduits de TVA actuellement en vigueur n'ont aucune incidence sur le prix TTC, donc aucune utilité. La deuxième objection concerne la directive européenne sur la TVA, mais dont il est sans doute possible d'utiliser les souplesses dérogatoires ou d'obtenir quelques révisions à la marge. La troisième objection est le coût budgétaire de telles mesures, mais ce manque à gagner ne pourrait-il pas être compensé, au moins partiellement, par l'instauration de droits d'accises sur certains produits de luxe ? Fiscalité et pouvoir d'achat étant intimement liés, ... Il faut conclure ! ... la modulation des taux de TVA est-elle une option envisageable par le Gouvernement ?

de nos concitoyens. Qu'il s'agisse des débats, des cahiers de doléances, des interrogations, des envois de courriers ou des contributions sur la plateforme, la question de la fiscalité est arrivée en premier. Évidemment, il y a beaucoup d'impôts en France, de nature très différente entre les ménages et les entreprises.

Nous devons effectivement répondre à cette baisse de la fiscalité souhaitée par nos compatriotes. La question est de savoir où, avec des comptes publics que vous savez dégradés. Il appartient au Président de la République de choisir les impôts qu'il proposera

Le grand débat, à mon sens réussi, apporte une preuve supplémentaire de la volonté des Français de participer à la décision publique.

délibérative », pour reprendre les termes de M. le Premier ministre. Le Sénat a fait, sous votre autorité, monsieur le président, dix propositions pour une démocratie plus participative renforçant la démocratie représentative et sans s'y substituer. Ces propositions portent sur le renforcement du référendum local, une rénovation du droit de pétition, à travers un droit de tirage citoyen, un droit d'initiative législative, un mécanisme de questions posées par des citoyens et, enfin, un assouplissement du référendum d'initiative partagée. Ma question porte sur ce dernier point : l'exécutif a-t-il le projet de reprendre la révision constitutionnelle ? Si oui, le fera-t-il par la voie parlementaire ? Proposerez-vous un nouveau texte ou comptez-vous sur le Parlement

allant vers davantage de démocratie participative, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Il me semble néanmoins que ce serait ne pas entendre ce qui a été dit dans le grand débat que de laisser les choses en l'état. Il appartiendra au Président de la République de préciser la manière dont il entend travailler sur ce sujet. En tout cas, et c'est essentiel, il ne s'agit absolument pas de substituer

Les Français ont ainsi appelé de leurs voeux une baisse massive de la fiscalité. Cette baisse devra concerner les particuliers autant que les entreprises, avec un objectif clair : augmenter le pouvoir d'achat de tous nos concitoyens. Cette baisse globale de la pression fiscale, pour concerner tous les Français, ne devra pas laisser de côté les outre-mer. Certes, des dispositions spécifiques existent déjà. Pourtant, elles se révèlent encore insuffisantes pour combler le différentiel de compétitivité de ces territoires par rapport à la métropole et à leur environnement géographique. géographique. Comment la baisse massive et rapide des impôts concernera-t-elle les outre-mer, notamment les entreprises ? Qu'est-ce que le Gouvernement prévoit d'apporter aux dispositifs existants, notamment pour ce qui concerne les TPE et les PME ? Le Gouvernement envisage-t-il d'élargir les aménagements fiscaux propres à certains secteurs d'activité à l'ensemble des entreprises ultramarines ?

de voir diminuer cette pression fiscale. C'est ce à quoi nous nous employons : nous avons comme objectif de diminuer le taux global de prélèvements obligatoires de 1 point de PIB à l'échelle du quinquennat. Cette baisse doit profiter à tous les territoires. Elle doit aussi être l'occasion d'améliorer la lisibilité de notre système fiscal. Nous aurons à travailler sur la fiscalité locale dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation ; ce sera très certainement l'occasion d'améliorer cette lisibilité. Nous aurons à travailler sur les impôts des ménages, comme sur ceux des entreprises. Vous savez les débats qui animent tant le Sénat que l'Assemblée nationale en matière de rationalisation des niches fiscales, de recherche d'économies et de lisibilité. Nous aurons à veiller à ce que les territoires ultramarins bénéficient, comme la métropole, des mêmes dispositifs d'exonération. La baisse de l'impôt sur les sociétés mise en oeuvre par le Gouvernement profite d'ailleurs à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur localisation.

quelles leçons tirez-vous du grand débat en matière de transition énergétique ? D'une part, la fiscalité écologique ne fonctionne qu'avec de la transparence, de la progressivité et de l'acceptabilité sociale. C'est d'ailleurs ce que le Sénat vous avait rappelé à la part, nos compatriotes attendent de la politique une réflexion sérieuse sur ce qu'on veut faire effectivement pour construire une écologie authentique. En guise de réponse, vous proposez une loi de programmation écologique qui serait soumise par voie de référendum. Quelle serait la question posée ? Faut-il, oui ou non, sauver la planète ? ... Nos politiques publiques environnementales manquent, depuis trop d'années, de cohérence et, surtout, de réalisme. Les Français ont le sentiment que les lois sur l'environnement, comme celle sur la transition énergétique de 2015, sont inconsistantes. Soit les objectifs sont fixés sur le très long terme et ne nous engagent pas réellement, soit ils le sont sur du très court terme et donc irréalistes, discréditant ainsi la parole publique. L'objectif intenable de 50 % de la part d'électricité issue du nucléaire d'ici à 2025 en est le meilleur exemple. Votre programmation pluriannuelle de l'énergie va d'ailleurs repousser l'échéance à 2035 et entrer ainsi en contradiction avec la loi de 2015. Nous attendons d'ailleurs toujours avec impatience le décret relatif

Enfin, ils n'opposent pas écologie et économie, écologie et solidarité, puisqu'ils pensent que les politiques écologiques peuvent leur permettre de réaliser des économies.

de 25 % en 2020, de 50 % en 2050, de sortie du glyphosate en trois ans, en accompagnant les filières. Les Français nous demandent d'agir au plan national et sur les territoires ; ils sont prêts à agir eux-mêmes.

Nos concitoyens savent bien que les services publics constituent le seul bien de ceux qui n'ont rien, et ils y sont légitimement très attachés. Aussi, quand l'école ferme, quand les options se réduisent comme peau de chagrin dans le lycée rural, quand les gendarmeries sont regroupées au chef-lieu de canton, quand l'hôpital public le plus proche est à plus d'une heure de route et que l'attente aux urgences peut durer des heures par manque de personnel, le sentiment d'abandon s'installe inexorablement, et c'est toute la perception d'appartenance à la communauté nationale qui se délite. Cette situation n'est évidemment pas brutalement apparue avec ce gouvernement, mais force est de constater son exacerbation ces derniers mois. Le numérique, s'il peut apporter des réponses partielles, ne sera jamais une solution globale et ne peut remplacer des agents compétents au contact des administrés. Comme l'a souligné le Défenseur des droits, il peut même, dans certaines circonstances, exacerber la fracture et le sentiment de relégation. Alors que la récente réforme de la justice éloigne le justiciable des lieux de justice, alors que la future loi pour l'école fait planer de lourdes hypothèques sur le maillage territorial du service public d'éducation, allez-vous faire évoluer la logique gouvernementale et tenir compte de l'attente de nos concitoyens, qui ne demandent pas une remise en cause de la fonction publique, mais des services publics, certes modernisés, parfois plus réactifs, bien présents à leurs côtés tant en milieu rural que dans les quartiers urbains ?

Nous avons comme objectif, avec Gérald Darmanin, de l'inverser en matière de finances publiques. Nous avons en tête que 1 200 points de contact ont été fermés en dix ans et que nous devons en réinstaller, peut-être en regroupant certaines fonctions support, mais en garantissant de la proximité, une présence physique sur le territoire.

Nous essayons d'apporter une réponse en termes de services publics sur chacun des territoires avec une présence humaine, en veillant à réformer aussi la manière dont nous gérons les femmes et les hommes qui servent l'intérêt général, les fonctionnaires, en les mettant au contact du public et en leur donnant ... Il faut conclure ! ... plus d'autonomie et de responsabilités au quotidien.

Cette responsabilité incombe à l'État et aux collectivités territoriales. Certes, nous avons fait des efforts, et la Cour des comptes a récemment noté que l'implantation des services publics dans les territoires ruraux résiste encore tant bien que mal, mais elle a aussi appelé l'État à améliorer la cohérence de ses services dans les territoires et à renforcer sa concertation avec les acteurs locaux. Il est évident que les récentes lois d'organisation territoriale n'ont pas vraiment clarifié le partage de responsabilité entre l'État et les collectivités. Dans nos travaux au Sénat, nous touchons du doigt cette réalité et en mesurons les effets délétères. Une partie du dynamisme et de la réactivité des pouvoirs publics locaux se perd inutilement dans les labyrinthes des circuits décisionnels. Pour corriger ces failles du maquis français, améliorer l'accès aux services publics, nous devons effacer les doublons, alléger les normes, libérer les initiatives.

des espaces de différenciation par lesquels les citoyens, les collectivités et l'État seront en mesure de construire une meilleure gouvernance de notre pays, du sommet à la base

présents d'une manière moderne sur les territoires. Nous savons bien que nous ne disposerons pas des services publics d'autrefois. Nous savons aussi que le numérique est un outil utile pour les services publics, mais que ceux-ci ne

Pour autant, impuissant face à cette crise, il a lancé son grand débat national. L'instrumentalisation des contributions le transforme en « grand bluff national ». En vingt-deux semaines, toutes les solutions n'émanant pas de l'Élysée ont été rejetées.

qui a prophétisé que « rien ne sera plus comme avant », ou va-t-il continuer à prendre et à imposer ses décisions seul ? Pour sortir de la crise, va-t-il enfin entendre la demande d'une grande conférence sociale, environnementale et territoriale associant l'ensemble des Français au travers de leurs représentants légitimes, à savoir les trois assemblées, les élus locaux, les partenaires sociaux et l'exécutif, afin que chacun prenne publiquement des engagements et s'y tienne

participé : un tiers par des contributions en ligne, un tiers dans 10 000 réunions partout sur le territoire et un tiers dans des cahiers citoyens. Nous pouvons bien sûr tous considérer que la parole de 1,5 million de personnes n'a pas d'importance, mais il me semble que cette parole a de la valeur et doit être entendue. Ce grand débat n'a pas opposé les Français et les corps intermédiaires : les organisations syndicales et patronales y ont beaucoup participé ; elles ont été incitées à produire des contributions. Nous avons monté des conférences nationales thématiques regroupant les organisations syndicales et patronales, les grandes associations, les associations

Pourtant, la plupart des Français sont particulièrement inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Plus personne n'ose dire aujourd'hui que l'école va bien. L'ascension sociale

Dans ce contexte difficile, à travers le déracinement des savoirs, le nivellement, la création des inégalités, l'école n'a plus d'identité et ne fait qu'aggraver les fractures territoriales, sociales et culturelles dans notre pays. L'école républicaine a cessé d'être nationale

appauvrissement intellectuel et cet abandon culturel produisent, dans un certain nombre de territoires et de quartiers laissés en marge, échec scolaire, violence, chômage, discrimination et un malaise dans lequel tant d'enseignants,

évoqué par nos concitoyens lors du grand débat. Je commencerai par saluer l'initiative de la ministre et du Premier ministre d'avoir lancé, dès octobre 2017, un plan pour l'accès aux soins.

des ARS, et ils seront impliqués dans les décisions de santé territoriales. C'est aujourd'hui le contrat que je veux conclure avec les citoyens : rien ne se fera sans les élus locaux. Je rencontre